reprenons si la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'l'intensification et l'extension du risque incendie dans la discussion des articles que nous ne sommes parvenus à l'amendement numéro 140 tendant à insérer un article additionnel après l'article 8.

Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de la commission. Comme certains autres. À la suite de discussions notamment avec le ministère parce que cet amendement vise à clarifier l'application des Zolder en cas de superposition entre des Zolder applicable aux infrastructures et des eaux des prévue par le code forestier. En effet, l'article L 134 14 prévoit qu'en cas de superposition des ALD. La mise en oeuvre de l'ensemble de ses obligations incombe au responsable des infrastructures pour ce qui les concerne. Cette règle, source de confusion tend donc à déresponsabiliser les propriétaires de construction sur leur propre terrain. Cet amendement vise donc à supprimer cette règle pour les voies ouvertes à la circulation publique et les voies ferrées tout en la maintenant pour les infrastructures de transport et distribution d'énergie au regard des spécificités techniques propres au Elder qui leur sont applicables. quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement, avis favorable du gouvernement. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté le 106 amendement du gouvernement Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. La réglementation des sites classés prévoit que les travaux et interventions dans les sites classés au titre du Patrimoine du paysage soient systématiquement soumis à une autorisation spéciale de travaux. Concrètement cela signifie pour le gestionnaire du site où le propriétaire, responsable de la réalisation des obligations légales de débroussaillement de devoir constituer un dossier de demande de travaux, ce dossier est ensuite instruit par l'inspecteur des sites soumis à avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites et l'autorisation est délivrée pour le ministre, vous conviendrez que cette procédure peut apparaître comme complexe pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement, censé se faire tous les ans et dans un délai maîtrisé à l'approche de l'été et donc de la saison des feux de forêt aussi cet amendement précise que les travaux de débroussaillement liés aux obligations légales de débroussaillement sont des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds au sens des réglementations relatives aux sites classés et aux abords des monuments historiques. Ce qui a pour conséquence de les dispenser de toute procédure au titre de ces mêmes réglementations toutefois le règle le gouvernement ne souhaite pas baisser d'autant la protection des sites à cette fin, l'abattage d'arbres de hautes tiges est susceptible, dans un certain nombre de cas de modifier l'aspect visuel des sites. Comme les sites sont souvent classés au titre de leur aspect paysager il est délicat de dispenser ses opérations impactantes de toute autorisation. C'est pourquoi l'amendement maintient une procédure d'autorisation, lorsque les obligations légales. Le débroussaillement conduisent à devoir couper des armes de haute tige mais prévoit qu'elle soit simplifiée et accélérée cette autorisation simplifiée et accélérée sera défini par décret. L'idée qui reste à définir complètement et de prendre une décision sur la base d'un court dossier de présentation, puis une réunion sur place entre le gestionnaire du site et l'inspecteur des sites au cours de laquelle les arbres à abattre seront marqués par cet amendement mesdames et messieurs les sénateurs. Le gouvernement espère être en mesure de simplifier et donc de mieux faire réaliser les obligations de débroussaillement je vous remercie. Merci madame la présidente. Il manquait quelques précisions rédactionnelles à la version initiale de cet amendement, le gouvernement ayant bien voulu apporter ces précisions. Ça sera un avis favorable d'autant plus que cet amendement vise à simplifier, comme l'a dit Madame la Ministre les eaux des dans des secteurs des des secteurs particulièrement protégés. Je vais donc mettre aux voix sa maman qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté le 142 monsieur le rapporteur. Oui merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à faire peser l'évacuation d'air émanant d'exploitation issus de la coupe de bois d'un propriétaire forestier sur la propriétaire de la parcelle. Sur le propriétaire de la parcelle, pardon. Dans le cas où cette parcelles se trouvent dans le périmètre où des eaux et des sont applicables. Pour résumer, quand un propriétaire a réalisé des Walder sur un terrain et sur le terrain voisin qui est forestier si le propriétaire de la Coupe fait une coupe il doit ça également s'occuper d'enlever les émanant de cette coupe. Quel est l'avis du gouvernement, avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté le 116 ans. Madame de Marco. Oui. Madame la présidente des obligations de débroussaillement sont fondamentales mental pour prévenir et limiter le risque incendie leur application, les moyens pour contrôler leur réalisations doivent être renforcés. Cependant, il est nécessaire d'atteindre le bon équilibre entre débroussaillement et préservation de la biodiversité. Ainsi le présent amendement propose de prendre en compte l'enjeu biodiversité dans les modalités de mise en oeuvre. Arrêté par les préfets. Un débroussaillement efficaces et compatible avec préservation de la biodiversité. Il suffit par exemple d'ajuster les périodes où sont réalisées ces débroussaillement en privilégiant l'Automne et l'hiver, on réduit l'impact sur la biodiversité. On réduit également le risque d'incendie puisqu'on limite les travaux forestiers, en saison estivale. Cet amendement répond également une préoccupation de la Fédération nationale des communes forestières. Il permet de renforcer la cohérence entre le code forestier, le code de l'environnement en matière de biodiversité. Selon les communes forestières. Ce manque de cohérence est actuellement un frein à la réalisation de nombreuses obligations des débroussaillement.

des eaux LD selon la nature du risque. Cet amendement vise à préciser que le préfet détermine les modalités de mise en oeuvre des Walder dans le respect de la biodiversité. Nous comprenons bien évidemment l'intention de l'amendement qui à l'image de plusieurs propositions que nous avons formulées dans le rapport. Et de l'amendement portant article additionnel que du monde adopter après l'article sept vise à une meilleure conciliation entre d'un côté la protection de la biodiversité et de l'autre la DFCI consultation. Conciliation que nous estimons non seulement indispensable mais surtout possible là dessus, nous serons d'accord. La rédaction proposée pourrait toutefois être source d'insécurité juridique pour les arrêtés préfectoraux LD. Ce n'est évidemment pas notre souhait le vôtre non plus j'imagine. Nous privilégions donc une solution qui s'appuieraient sur une instruction technique adressée aux préfets afin de clarifier le droit existant pour trouver des solutions en cas de conflit entre la défense des forêts contre l'incendie et la protection de la biodiversité. C'était le sens de la recommandation numéro 43 d'ailleurs de notre rapport d'août 2022. C'est la raison pour laquelle nous mais émettront un avis défavorable sur votre amendement madame Di Marco. Madame la Ministre, quel est votre avis. il n'y a pas lieu d'après nous de subordonner le code forestier au code de l'environnement comme vous le proposez ce d'autant plus en visant l'article L 110 tirer 1. Du code de l'environnement qui est un article très général sur le respect des milieux et de la biodiversité en général certes quand on défriche, on enlève des végétaux, mais les objectifs de sécurité publique doivent primer dès lors qu'il ne s'agit pas d'espèces ou d'habitat protéger spécifiquement à cet effet les 2 réglementation sur la biodiversité Elder doivent s'articuler et aucune. N'est subordonnée à l'autre. Nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable Merci madame la présidente, j'ai écouté avec grande attention à notre collègue était Marco. Je suis un peu surprise. Ma chère collègue que. Lorsqu'on parle d'des vous voulez débroussailler ça débroussailler c'est comme s'il y a quelques jours des fêtes de Pâques, vous voulez faire d'omelette Pascale à cinq sans casser les oeufs. Madame de Marco. Comment. Je je relèverai pas la remarque en réalité c'était très simple, c'était éviter certaines périodes. Mais j'ai été convaincu par vos arguments, je vais retirer. Merci. 2 amendements en discussion commune le 141 monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de la commission vise à créer autour des campings. Une zone d'LD de d'obligation légale de débroussaillement de 50 mètres, voire même de 100 mètres sur la volonté des maires. Attendez, madame la ministre, avant que vous donniez votre avis je donne la parole à Madame Pentel pour le 84. Il y en a 2. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à lever certaines ambiguïtés, concernant la responsabilité de chaque propriétaire hors zone urbaine, le propriétaire de chaque construction est tenu de débroussailler dans un rayon de 50 mètres. Cette zone est susceptible de dépasser les limites de propriétés notamment quand le propriétaire voisin n'a pas de construction dans le périmètre de 50 mètres. Le propriétaire de la parcelle doit être identifié par l'intervenant et une demande d'intervention doit être adressé par courrier recommandé avec accusé réception. Il revient paradoxalement à la personne responsable de l'eau et le D de demander au cadastre à qui appartiennent les parcelles pour demander l'autorisation d'intervenir, ce qui ouvre des possibilités de contentieux non négligeables. Par ailleurs, de fait, les propriétaires des petits se trouvent désavantagés par rapport aux propriétaires de grandes parcelles aussi cet amendement propose de mieux identifier le principe selon lequel chacun doit contribuer à remplir ses obligations à proportion des pincettes dont il est propriétaire. Je vous remercie. Si monsieur le rapporteur. Quel est votre avis sur cet amendement madame Platel vient de nous présenter. Merci madame la présidente. Donc c'est monsieur Roux qui avait posé cet amendement le code forestier prévoit que les travaux au LD sont à la charge du propriétaire de la construction chantiers ou installations ou du propriétaire du terrain, selon la nature des obligations. Il ne semble pas pertinent de modifier cette distinction comme le propose cet amendement qui aurait pour conséquence de déresponsabiliser les propriétaires occupants ou bailleurs des constructions chantier ou installation ça sera donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Madame la Ministre, quel est votre avis sur. Ces deux amendements. Le même que monsieur le rapporteur. Donc sur le 141. Avis favorable et une demande de. Retrait pour le 84 sinon avis défavorable. Madame Pentel voulait dire quelque chose. Notre merci. Donc je mette au mais on voit le 141 qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté. Et il fait tomber le suivant. Nous Nous passons maintenant aux 2 au 65 qu'ne présente Madame Jourda. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à créer un nouveau document unique, Claire et facilement identifiable à destination des particuliers pour s'assurer de la bonne réalisation des aux Nous estimons en effet comme propriétaire de terrain. Soumis à une obligation légale de débroussaillement devrait pouvoir obtenir un document clair rappelant les informations relatives à la situation de leur terrain et en conséquence, la nature des obligations qui leur incombent et les mesures qui doivent être prises pour y répondre. Actuellement, aucun document spécifique n'existe. L'article 11 de la proposition de loi prévoit ainsi dans un cas la remise d'une attestation de conformité, puis dans un autre une attestation sur l'honneur. Nous proposons donc par cet amendement. La création d'un diagnostic de l'obligation légale de débroussaillement d'Old qui seraient établis à titre gracieux par l'entrepreneur de travaux forestiers certifiés ayant réalisé les travaux de débroussaillement il deviendrait ainsi. Le document de référence en matière d'elle le des si nous souhaitons que figure dans la loi. Certaines des informations donc devront comprendre ce document. Nous pensons néanmoins nécessaire de renvoyer à un décret sa mise en oeuvre. Merci. Non madame var, alias Monsieur Guey, pardon. Merci madame la présidente madame Nice, mes chers collègues. On a le même amendement. J'ajoute que nous pensons que ça serait utile en cas de vente notamment et et de l'acquisition d'un terrain par un nouveau propriétaire pour que ce propriétaire soit informé de ses obligations. De comment le faire et donc nous pensons que nos deux amendements nous amendements communs vont plutôt dans le bon sens et dans cette proposition de loi, je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission. Merci madame la présidente. Sur ces deux amendements présentés par Madame Jourda et et Monsieur Gay. Ça sera un, un, une demande de retrait on avis favorable. Pour une raison c'est qu'on considère que ces amendements sont satisfaits car ils reprennent avec un vocable différent l'idée d'une attestation de conformité des Walder. Ce que nous avons prévu un petit peu plus tard dans l'article 11. Fait pour le gouvernement sur les 65 comme sur le 92. Le gouvernement émet un avis demande le retrait sinon un avis défavorable.

Il n'est pas adopté sur le 92 même vote. À l'article 9, un amendement numéro 75 qui est présenté, toujours pas Madame Jourda. On On vient de passer à l'article 9 et on a l'amendement 75. En tout cas en ce qui me concerne et donc un amendement qui Madame Jourda homme madame Marie baie où Monsieur Gillet. Cet amendement vise à consacrer dans la loi la possibilité pour les maires et non l'obligation de pouvoir organiser une m'utilisation des eaux elle des des particuliers. Actuellement, certaines communes procède déjà à la réalisation des elle le des. À la charge financière bien évidemment des particuliers concernés. Dans un souci d'efficience cet amendement propose de reconnaître aux communes la possibilité de mutualiser ce type d'action entre plusieurs particuliers cette possibilité aura 3 bénéfice d'une part, elle permettra à une commune de s'assurer que l'ensemble des eaux elle le des sur son territoire a été réalisée. D'autre part, elle lui permettra de pouvoir faire des économies d'échelle en négociant des prix attractifs avec les entreprises, en charge du débroussaillement

et moi je vous. Défendent de 75. Le 75. Et tu vise à créer un diagnostic de l'obligation légale de débroussaillement. Oui alors comme c'était un amendement de coordination. C'est bien d'ailleurs ce que je pensais au départ ils tombent puisque le le l'amendement précédent précédent de mandat un diagnostic au LED a été. je mets aux voix l'article 9 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté l'amendement. Nous prenons maintenant 2 amendements identiques, on commence par le C'est à vous. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées. Tu es la main demain que je souhaite présenter qui est co-signé par très nombreux collègues. Oui merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur ces deux amendements qui parce que notre chère collègue le sénateur Burgos a bien voulu modifier le sien deviennent complètement identiques, je vous deux donnerai donc un avis favorable sur ces deux amendements. Madame la Ministre, quel est votre avis sur ces deux amendements identiques, avis favorable quand le monsieur le rapporteur. D'accord très bien. Je vais donc mettre aux voix. Ces amendements identiques. Favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils sont adoptés madame Jourdain, nous voilà au 66. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a été défendu. Il a été les fans du mal. La primaire. Pire que tout le monde a bien suivi tout à l'heure. Donc quel élève. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Merci madame la présidente. L'article L 131 14 du code forestier permet déjà. Madame Jourdain aux collectivités territoriales de faire les Walder à la place des particuliers et à leur demande. Dans ce cas, il est prévu qu'elle se fasse rembourser les Walder par c'est particulier l'amendement est donc partiellement satisfait. Si l'idée de l'amendement et d'aller plus loin pour tendre vers une forme de service public des eaux ALD sous l'égide des collectivités territoriales, nous n'y sommes pas favorables, en tout cas pas comme l'amendement le formule et de ce qu'on a pu entendre les communes elles-mêmes n'y sont pas favorables. En effet la notion de mutualisation des travaux et vague surtout l'amendement ne précise pas sûr qu'qui serait imputé la charge de ces travaux. La mutualisation des Zolder implique-t-elle une taxe. C'est pour ça que nous vous demandons de retirer votre amendement à défaut ça sera un avis favorable. Madame la ministre. À vie. Demande de retrait sinon avis défavorable exactement les mêmes raisons. Monsieur le rapporteur. Madame Jourdain. Explications de vote. Explications de vote et tout simplement je vais retirer cet amendement peu Compte-tenu. Des explications qui viennent d'être donnés. Mais je tiens quand même à dire que la mutualisation de ce type de travaux bien entendu réalisés par les collectivités locales auraient été imputée au propriétaire des des qui n'auraient pas souscrit aux travaux de d'obligation de débroussaillement, c'était tout à fait clair dans l'amendement présenté. Le 70, madame Ribet. Alors messieurs les rapporteurs si madame la un porteur si les communes peuvent déjà mutualisé nous il nous semble par cet amendement important de préciser les modalités de remboursement des frais engagés par les communes et leurs groupements où les syndicats compétent lorsqu'elles procèdent. Aux opérations de débroussaillement. Et c'est l'objectif de cet amendement. Quel est l'avis de la commission. Montrer que il serait prévu alors déjà à la base dans le code forestier, il est prévu que les collectivités territoriales comme j'ai dit juste avant puisse déjà. Réalisé les ALD à la place des particuliers à leur demande. Par contre cet amendement viendrait remplacer. La formulation actuelle du remboursement des frais engagés. Pour préciser que la prise en charge et Zolder donnerait lieu au paiement d'une redevance par leurs propriétaires concernés et que le montant de cette redevance serait fixé par décret. Nous préférons au niveau de la Commission rester sur le droit existant, une convention de réalisation des Zolder, à la place des propriétaires, les modalités de remboursement on passa au conseil municipal, c'est plus clair, c'est plus libre et on n'est pas sur une redevance obligatoire. Oui donc ça sera une demande de retrait ou un avis défavorable, Le Gouvernement émet le même avis parce que compte tenu de la diversité des situations et donc des coûts des travaux très divers, il faut rester remboursement au réel du coup effectif des travaux, comme le prévoit la loi actuellement car il sera impossible de. Ce montant de redevance selon un barème national par décret. Bon pour ces raisons, on vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Je vais donc madame Harribey pour une explication de vote. Oui, nous il nous semble que c'est important de d'avoir un barème parce que très souvent, les communes n'ayant pas là une base juridique suffisante abandonne. Le système de la redevance et donc le système de de la de de débroussaillement pour le compte des particuliers. Donc on maintient la maman. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté le 144 monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article L 135 2 du code forestier prévoit qu'en cas de violation constatée du Noël Le maire ou le cas échéant le préfet met en demeure la personne de réaliser ça doit aider. Par contre si malgré cette mise en demeure la personne ne réalise toujours pas ses Walder. Il faut que le maire saisissent le préfet qui peut alors prononcer une amende administrative cet amendement vise à simplifier. La mesure et faire en sorte que sans que le maire sera obligé de saisir le préfet, le préfet de lui même peut. Prononcer une amende administrative. Quel est l'avis du gouvernement. Cette simplification devrait permettre une meilleure mise en application de l'article L 135 de du code forestier, l'avis du gouvernement et donc favorable. Merci madame la présidente. Merci je mais on voit cet amendement lui favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Je vais mettre aux voix maintenant. L'article 9 bis qui et pour qui est contre qui s'abstient adopté. À l'article 10 l'amendement 39 monsieur Denis Colin. Il a, j'ai trois amendements, madame la présidente. Vous voulez que j'ai présente les 3 ensemble volontiers si. Militant. Donc le premier amendement cet amendement vise à étendre également l'application du crédit d'impôt aux travaux débroussaillement réalisée par un groupement forestier et visées par le code forestier pour les petites parcelles il y a souvent, souvent, les propriétaires qui se mettent un groupement pour permettre de d'être plus efficace. Le 2ème amendement concerne les travaux de débroussaillement aussi qui sont souvent réalisés par les propriétaires eux-mêmes or ces travaux réalisés dans le but de limiter la propagation des incendies ont un but d'intérêt général. Il convient donc d'étendre le crédit d'impôt aux travaux réalisés par les propriétaires n'ayant pas recours à un prestataire pour leur réalisation. Et le 3ème amendement c'est dans dans dans un souci d'harmonisation avec le défi forestier cet amendement vise à tenir compte de la situation de famille pour la détermination du crédit d'impôt. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements. Merci madame la présidente. Alors sur ces trois amendements, le premier de monsieur. De Nicolay. Le 39 rectifier ça sera un avis défavorable sur cet amendement, cher collègue. Il ne me semble pas important opportun détende, le bénéfice de ce crédit d'impôt aux groupements forestiers pour plusieurs raisons, premièrement votre amendement va selon moi l'encontre de l'ambition initiale de ce crédit d'impôt. Notre but est plutôt de cibler les personnes physiques qui, faute de ressources suffisantes, ne sont pas en mesure de réaliser les ALD par leurs propres moyens. Les groupements forestiers se constituer en vue d'une exploitation de la forêt et les revenus qu'ils tirent de cette exploitation devrait légitimement servir à financer ces dépenses de réalisation des ALD. De plus les membres d'un groupement forestier bénéficient déjà de plusieurs mécanismes de réduction et d'abattement d'impôts donc il ne nous semble pas opportun de les inclure dans ce dispositif spécifique aux zoo LD. Concernant le 40. Rectifier toujours de notre collègue de Nicolet. Un avis défavorable également. Il va selon moi à l'encontre de l'intention initiale de la proposition de loi qui vise à inciter les particuliers à recourir à des professionnels certifiés et encourager le développement d'une économie des ALD. Par ailleurs, le dispositif que vous proposez serait difficile à contrôler par l'administration fiscale. Puisque la condition d'attribution de ces crédits d'impôt reposerait uniquement sur une déclaration de bonne foi du bénéficiaire. Ce mécanisme conduira nécessairement à des abus. également un avis défavorable. Vous m'en pardonnerez chers collègues sur le 3ème amendement le 49 rectifié. Un avis défavorable qui introduit une différence de traitement injustifiée entre les personnes célibataires. Les personnes mariées ou pacsées. Le coût des opérations débroussaillement ne ne varie pas lui selon la situation familiale. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une telle distinction. Merci. Si, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame. La présidente. Monsieur le sénateur, de qui. En fait pour les trois, que ce soit le 39 le. 40. Et le 49. Ratifier le gouvernement souhaite rappeler qu'il n'est pas envisageable de créer, comme le propose cet article un crédit d'impôt mécanisme qui vivent à inciter un comportement. Donc un crédit d'impôt en faveur de dépenses dont la réalisation résulte d'une obligation légale. Dès lors, il est difficilement concevable d'en étendre la portée et donc le coût qui est supportée par la puissance publique. Par ailleurs les mesures fiscales ont vocation à être discuté en projet de loi de finances.

de ces parcelles donc. Évidemment. Si ici uniquement le le le le propriétaire qui a quelques fois très âgés ne peut pas le faire et c'est dommage que les groupements forestiers ne puisse pas en bénéficier mais enfin c'est votre position. le dernier amendement sur le défi forestier c'est simplement. Le défi Forestier tient compte de la situation familiale. C'était pour appliquer la même chose. Dans le cadre de de de ce débroussaillement de pour la lutte pour les incendies, pour être en cohérence. Ouais, c'est simplement ça. Mais je maintiens les amendements.

Même vote 49 même vote même vote aucun être adopté je mets souvent maintenant. L'article 10 ce qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adoptée après l'article 10. Monsieur de Nicolas il vous avez la parole pour le l'amendement 41. Les choses s'enchaînent. Donc le, l'article 41, cet amendement vise à créer un crédit d'impôt pour l'aménagement de points d'accès à l'eau stabilisation et de retournement accessibles, notamment pour les véhicules de lutte contre les incendies et lorsque ce point d'eau peut être utilisée pour protéger une habitation. C'est le premier amendement. Vous voulez que je dise il a aime ou le respect de l'obligation légale de débroussaillement certains dispositifs d'autoprotection, ça vire ainsi efficace pour protéger les habitations. À ce titre, le fait d'équiper une piscine ou une citerne d'eau d'une mono moto-pompe un. Heure peut être utilisée pour arroser une habitation et ainsi la protéger des les incendies et décharger hein oh d'autant les sapeurs-pompiers de plus ce dispositif de protection de l'. Permet comme indiqué dans le rapport ci-dessus de libérer un camion de sapeurs-pompiers pour contenir le feu ailleurs et donc cet amendement vise donc à inciter les particuliers à s'équiper de dispositifs d'autoprotection en créant un crédit d'impôt s'appliquant aux dépenses d'acquisition de ceux-ci. Six, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Merci madame la présidente. Ça sera le même avis sur les deux amendements présentés par notre collègue de Nicolet. Pour les mêmes raisons, donc je l'ai, je les je les citerai qu'une seule fois je me répéterai pas. On va gagner du temps. Premièrement. Le crédit d'impôt qui a été mise en place de sur la volonté de la mise en place de ce crédit d'impôt au niveau de la PPL, c'est uniquement pour la nécessité de créer une incitation vers les particuliers. À réaliser leurs Zolder dans un contexte d'une très faible, réalisation Elder dont notamment le coût peut être particulièrement prohibitif unifie prohibitifs pour les particuliers. Donc on s'adresse aux particuliers et uniquement pour les Zolder et donc on ne voit pas l'opportunité de multiplier les crédits d'impôts dans cette PPL donc ça sera une demande de retrait sur les deux amendements ou un avis défavorable. Merci madame la ministre. mais en complément. Vous dire simplement que la mesure proposée qui constitue une nouvelle dépense fiscale n'a fait l'objet d'aucune évaluation de chiffrage préalables les mesures fiscales comme je vous l'ai dit tout à l'heure ont vocation à être discuté en projet de loi de finances et donc je vous engage. a envisagé cette cet amendement plutôt dans ce cadre, donc je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et sinon on ne le gouvernement émet un avis défavorable. Ils sont retirés, me dit l'auteur des amendements et nous passons donc aux 91 madame Maria. Les obligations légales de de débroussaillement figure en bonne place des responsabilités qu'assument les mères, comme le souligne la Fédération nationale des communes forestières une simplification une harmonisation et un plus grand soutien de l'État sont attendus pour accroître l'application de cette règle réglementation qui reste moyen efficace pour se protéger du feu dans ce cadre, il faut rappeler que les collectivités aussi ont besoin d'être soutenus pour la réalisation de leur LD une commune rurale qui a un grand linéaire de route et un budget bien évidemment en lien avec sa population peut difficilement réaliser les Walder sur son territoire sans accompagnement face à la récurrence du risque incendie et la progression de la forêt dans certains territoires. Il est impératif que le gouvernement réfléchisse aux dispositifs d'accompagnement et d'aide financière qui pourrait être mises en oeuvre pour aider les les communes à faire face à ces. madame Jourdain. Président. Mes chers collègues. Cet amendement vise à soulever une problématique importante à l'heure où les finances et les marges de manoeuvre des collectivités territoriales sont plus que jamais contrainte et ce particulièrement en zone rurale. Nous demandons ainsi la remise de d'un rapport du gouvernement au Parlement, visant à réfléchir aux dispositifs d'accompagnement et d'aide financière qui pourraient être mises en oeuvre pour aider les communes à faire face à leurs obligations légales de débroussaillement face à la récurrence du risque incendie et la progression de la forêt d'un certain territoire certaines communes rurales avec peu de moyens, dans des zones très forestière se retrouvent en effet démunies financièrement pour réaliser leurs au Il s'agit notamment des communes avec un Graal linéaires de route et un budget très restreint du fait d'une population très faible, certains territoires très forestiers sont ainsi particulièrement concernés comme dans les Cévennes. Or de solutions existent. Face à ces situation soit nous réduisons les obligations des communes, un terme doit le des. Ce que nous ne souhaitons pas, soit nous réfléchissons à la mise en place de dispositifs d'accompagnement spécifique pour les communes hein difficulté c'est l'objet du présent amendement. Six, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Merci madame la présidente, concernant ces deux amendements de nos collègues Madame Breillat c'est Madame Jourda. Et n'étant pas favorable dans cette PPL à introduire des demandes de rapport, ça sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la Ministre même avis même avis. Je vais donc mettre aux voix l'amendement d'abord 91 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté sur le 64 même vote même vote il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 11 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement numéro de monsieur Burgot. Merci beaucoup madame la présidente, madame la ministre, Madame et messieurs les rapporteurs. Afin de faciliter l'application du régime de la gestion d'affaires et de manière subsidier de l'enrichissement injustifié. Cet amendement propose d'introduire un nouvel article dans le code forestier. Cet article précise que l'indemnisation d'une personnes qui se substitue aux titulaires défaillant d'une obligation légale de débroussaillage suit des règles de la responsabilité quasi contractuelle prévue par le code civil. Ces dispositions crée également une présomption d'égal sur la base de laquelle, d'une part le débroussaillant serait réputé être accomplie dans l'intérêt du titulaire défaillant et d'autre part que l'économie que ce dernier réalise serait réputée constitue un enrichissement au sens des dispositions du code civil, il s'agit à l'espèce de permettre d'indemniser les personnes qui se substituer leurs voisins défaillant pour assurer les obligations de débroussaillage qui lui incombe. Telle est l'amendement proposé et co-signée par de très nombreux collègues. Merci. Que de la ville. Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Merci madame la présidente. Chers collègues comme vous, nous vous l'avions dit en commission. Il nous est difficile d'évaluer à ce stade les tenants et aboutissants de cette proposition notamment d'un point de vue juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de redéposer cet amendement en séance dans le but de recueillir l'avis du gouvernement sur cette proposition. Et donc notre avis c'est à vie du gouvernement. Merci.

qu'une personne puisse se se substitue aux titulaire défaillant d'une obligation légale de débroussaillement. Seules des personnes morales communes ou États peuvent le faire au titre du code forestier actuel la substitution pour des motifs certes légitime que vous évoquez, me semble de nature à créer de la complexité dans les relations de voisinage, voire un risque d'engorgement des tribunaux. Dans ces conditions. Nous vous demandons de bien vouloir accepter de retirer votre amendement. À défaut, notre avis est défavorable. Et c'est donc maintenant l'avis du rapporteur. Oui madame la présidente, nous nous rangeront derrière l'avis du gouvernement, donc un avis défavorable. Monsieur Burgot. Merci à la. Écoutez, j'ai écouté l'avis de la ministre de monsieur le rapporteur. Mais pour une fois je vais être un peu moins sage Madame la Ministre parce que je ne pense pas que cet amendement a d'abord créer un article complémentaire, il est pas dans le code forestier et puis je suis pas sûr qu'on avait un amant engorgent. Plus. Les juridictions donc je le maintiens et je m'en remets à la sagesse du Sénat. Très bien je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement 23, madame la présidente Delattre. Merci madame la présidente, mes chers collègues au regard du risque feu de forêt l'installation d'une construction quelle que soit sa nature, au sein du massif forestier entraîne une aggravation du risque en terme d'aléas et peu dénaturer la physionomie d'un territoire et son organisation en terme de défense incendie. Il est donc impératif que tout projet qui seraient autorisés au contact des espaces forestiers doivent proposer une véritable stratégie de mise en sécurité par rapport risque incendies de forêt pour être compatible avec son site d'implantation en ce sens le code forestier dispose que dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendie de forêt toute opération de nouvel aménagement. Comporte dans son périmètre une bande de terrains non bâtis à maintenir en état débroussailler d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres isolant les bois et forêts, des constructions en vue de satisfaire leurs obligations légales de débroussaillement les promoteurs de ces opérations d'aménagement pourrait solliciter l'accord des propriétaires forestiers. Forestiers pardon voisin pour réaliser des travaux de défrichement et la création d'une bande inconstructible sur leur terrain voisin. L'objectif de cet amendement certainement ambitieux et de rendre obligatoire la bande inconstructible dans le périmètre du projet de construction. Je vous remercie monsieur le rapporteur. Merci madame la la présidente. Cher collègue Nathalie Delattre. Je le dis avec beaucoup de bienveillance mais votre amendement mélange à mon sens de sujet. Les, des, d'une part et la maîtrise de l'urbanisation dans les zones particulièrement à risque. D'autre part. Au titre des ALD. Vous savez qu'il existe déjà une obligation débroussaillement autour des constructions d'au moins 50 mètres ou au plus de 200 mètres sur ce point, l'amendement est satisfait. L'amende votre amendement propose-lui par ailleurs de prévoir une interdiction totale de construction dans cette bande péri Métral. C'est déjà l'objet des PPRI Arif et des documents d'urbanisme. En tout état de cause une interdiction générale de construction semble semble non proportionnée de plus des interdictions auraient sans doute plus de sens dans des zones éloignées de toute construction au coeur même des massifs, par exemple, ça sera donc soit une demande de retrait soit un avis défavorable Merci madame la présidente, madame la sénatrice de la alors. Cet amendement s'appliqueraient indifféremment à une multitude de situations différentes. Ce qui d'après nous, n'est pas souhaitable en effet les zones particulièrement exposées au risque d'incendie sont déjà inconstructible au titre du code de l'urbanisme, en application de l'article L 111 tirer de de plus permettent que le PLU les ouvre à l'urbanisation serait commettre une erreur manifeste d'appréciation. Il n'améliore donc pas la prise en compte dans le droit de l'urbanisme, des risques d'incendie sur les constructions nouvelles en cohérence avec la volonté du Sénat de davantage intégrer le danger de feux de forêt dans l'urbanisme, le gouvernement propose un dispositif consistant à élaborer une carte nationale caractérisant la susceptibilité du territoire au danger prévisible de feux de forêt et de végétation en complément de cette mesure, le gouvernement serait favorable à la mise en place d'un dispositif nouveau qui permettrait, sur la base des zones délimitées par cette carte la mise en place d'une servitude d'utilité publique par une procédure simplifiée, comparativement à celles d'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie et et de forêts cette servitude permettrait de s'opposer à de telles constructions ou de leur imposer des prescriptions. Ce qui va dans le sens de votre amendement et c'est tout le sens de notre amendement numéro 109 déposée par le gouvernement, je souhaite si vous le voulez bien, que vous retirez votre amendement sinon nous émettrons un avis défavorable je vous remercie. donc. Pardon. Nous passons donc maintenant à l'amendement 67 de Madame Jourda. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement étonnamment demande d'appel qui vise à tirer un bilan du naissent de l'expérimentation menée en Occitanie par l'Union régionale des collectivités forestières Lur confort met ainsi à disposition des communes. Un outil cartographique permettant à chaque citoyen de connaître ses obligations en terme d'obligation légale de débroussaillement. Une fois de plus notre souhait devrait au maximum à la sensibilisation et à la mise en place d'une pédagogie en matière de OL des pour que tous les particuliers bien connaissance de la loi de leurs obligations et également de l'intérêt de réaliser ses travaux en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Il s'agit également dans le cas présent d'apporter un appui à des communes qui parfois sont démunis ah matière le des. Sur la base de ce bilan qui se traduirait donc par la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an nous pourrions ainsi déterminer si l'action menée en Occitanie méritent d'être généralisés sur l'ensemble du territoire français ou si les spécificités de chaque territoire ne rein de pas pertinent. Merci madame la présidente. Concernant cet amendement de notre collègue Gisèle Jourda. Alors déjà c'est une demande de rapport, donc vous connaissez notre vision sur les rapports mais. J'irai plus loin. Ça sera une demande de retrait. Un avis défavorable notamment pour une raison, c'est que les conclusions de cette étude et le rapport sur ce qui est fait, notamment en Occitanie. Finalement les anticiper puisque dans l'article 8, on a décidé une inscription des ALD dans les documents d'urbanisme, ce qui permettra d'informer directement. Chaque habitant de sa situation par rapport aux zoo donc la réponse ayant été devancée. Nous vous demandons de retirer votre amendement sinon ça sera un, avoir un avis défavorable. Non non ne mettez. Et entendu donc ceux-ci je le retire. J'ai dit que c'était un amendement d'appel mais je ne souhaiterais pas que les travaux mis en oeuvre donc au niveau de l'Occitanie au plan régional tombent dans les oubliettes, comme c'est souvent le cas et on passe souvent à côté de vraies solutions. Merci l'amendement 110 Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Nous partageons l'esprit des articles 12 et 13. Issu des travaux de la commission spéciale et souhaitons leur apporter des précisions. Nous sommes attachés à fixer les priorités d'action en fonction des contextes territoriaux et en concertation avec les maires. C'est pourquoi fixer une liste contraignante de communes à doter de plans de prévention des risques d'incendie de forêt ne nous semble pas souhaitable. Nous proposons plutôt d'établir une liste de communes exposées à un danger de feux de forêt élevé sur la base d'une carte établie sous la responsabilité de l'État. Nous avons aussi fait notre l'idée d'une procédure de modification simplifiée des plans de prévention des risques d'incendies de forêt, nous souhaitons renforcer la sécurité juridique de cette procédure et limiter les contraintes d'évaluation environnementale. La modification simplifiée permettra ainsi de modifier ses plans en 4 à 6 mois au lieu de 18 mois actuellement avec cet amendement, l'État pourra réagir plus vite après que les maires et réaliser les travaux de protection. C'est pourquoi nous espérons un accueil favorable de cet amendement. Merci. Merci madame la présidente. Nous donnerons un avis favorable à l'amendement du gouvernement sous réserve. De l'adoption de ce sous-amendement. Qui vise à main. Tenir l'identification par arrêté d'une liste de communes où la protection contre les incendies rend nécessaire la dans l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels. L'adoption de l'amendement du gouvernement conduirait en effet à supprimer cette partie de l'article 12. Ce qui serait contraire à l'intention des auteurs de la proposition de loi et aux orientations de la Commission par ailleurs ce sous-amendement conserve les précisions apportées par l'amendement du gouvernement. Concernant la procédure de modification simplifiée des pépés R. I. F en lui apportant des clarifications rédactionnelle. Madame la Ministre quel est votre avis sur le sous-amendement de la commission. d'un plan de prévention des risques d'incendie, plutôt que la voie de compromis qui a souhaité proposer le gouvernement sur ce point. Nous prenons acte de votre position que traduit votre amendement. La suite de votre amendement fiabiliser la rédaction. Que nous avons proposé en reprenant l'esprit des travaux de la commission spéciale il précise ainsi la procédure de modification simplifiée des plans de prévention des risques d'incendie. Je me réjouis que sur ce point nous habitue si on a une mesure opérante et pragmatique au bénéfice des acteurs de terrain, c'est pourquoi nous nous en remettons à la sagesse du Sénat. Monsieur le rapporteur. Bien je vais donc mettre aux voix le sous-amendement 150 qui a reçu un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté, je mets maintenant aux voix. L'amendement du gouvernement. Ainsi sous-amendé qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Je me vois l'article 12 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté l'article 13, une demande de parole de monsieur Cette prise de parole. À propos d'un amendement qui a été retiré en commission qui visait à à créer un article additionnel à l'article 13 et portant sur. La nécessaire signalétique des élus en présence d'événements et et d'incendie pour pouvoir mieux effectivement les repérer, sachant que l'ensemble des autres acteurs dispose d'éléments de signalétique important je voulais Madame la Ministre, attirer votre attention cet amendement a été retiré parce que c'était de l'or du règlement et non pas législatif néanmoins c'est une demande forte des élus de pouvoir disposer d'une signalétique leur permettant d'être identifié sur les moments effectivement de crise sur les moments d'incendie. Donc je voulais vous le signaler et il serait souhaitable qu'on puisse trouver une solution à ce niveau-là, je vous remercie. Madame la Ministre l'amendement 109. Nous retirons l'amendement 109. Très bien. Le 21, madame la présidente Delattre. Monsieur Cabanel, merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Les chambres d'agriculture connaissent parfaitement les caractéristiques, les problématiques et bien évidemment, les risques de leur territoire. Cette expertise. Nous sommes le précieuses il serait nécessaire de valoriser et de s'en servir c'est pourquoi cet amendement vise à inclure et charmeur agriculture dans l'élaboration, à destination des communes une une carte d'aléa permettant de cartographier le risque dès samedi 2. De surfaces agricoles et de végétation. Ils sont séparés donc. Madame, monsieur, ne le rapporteur. Quel est votre avis sur l'amendement que monsieur Cabanel, vient de présenter le 21. Merci madame la présidente. Commentaire de de la commission sur cet amendement. On, on voit mal. Très concrètement pourquoi la chambre départementale d'agriculture serait spécifiquement consulter sur la réalisation de ces cartes d'aléas. Alors que l'article 13 ne prévoit à ce stade aucune autre forme de consultation. Par ailleurs il serait pour le moins surprenant de prévoir dans une loi une consultation des directions départementales des territoires qui relève de l'autorité du préfet. Pour ces raisons, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Madame la Ministre même avis. Merci.

Alors cet, cet amendement est un un amendement d'un tout petit peu de précisions sur le fait de, de la communication d'une carte graphique des aléas. Qui pourraient se. Difficile à appréhender pour les communes regroupements de communes, et donc il est important qu'elle dispose d'éléments d'appréciation explicative pour c'est pour qu'elle puisse prendre les décisions adaptées. Donc c'est pour préciser un peu plus le l'article l'alinéa 4 de l'article 13. La commission. Merci madame la présidente. Il ne nous semble pas nécessaire de prévoir une transmission des critères d'appréciation des cartes d'aléas prévue à l'article 13, une méthode d'élaboration de ces cartes seraient élaboré au niveau central et devrait être partagée pour l'information de toutes et tous. Mais une transmission systématique de cette méthode aux élus locaux ne semble pas nécessaire cette transmission peut au demeurant, se faire sans que la loi n'est à le préciser. Vous l'aurez compris, il s'agit de vous proposer une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable à la main ministre même avis absolument. Nous passons maintenant à l'amendement 11 monsieur Burgot. Merci madame la présidente. Mes chers collègues. Afin d'être opérationnel. La carte ah d'aléas doit être une cohérence avec le le périmètre des terrains soumis à des obligations de débroussaillement. Elle devra aussi faire l'objet d'une concertation avec les SDIS particulièrement concernés. Telle est l'objet de cet amendement qui concourt à une meilleure préparation de crise ainsi qu'à la planification des moyens à déployer. Cet amendement fait écho à notre amendement numéro 98. Dans je lui prédis pas un grand avenir mais néanmoins comme pour la cartographie des Walder annexé aux différents documents d'urbanisme, la carte d'aléa pour être fonctionnel doit être en cohérence avec le périmètre des terrains soumis à des obligations de de débroussaillement. Elle devra aussi faire l'objet d'une concertation avec les. Particulièrement concernés. Je répète que la prévention est un sujet impliquant une multitude d'acteurs, nous sommes convaincus du fait qu'il est à ce titre nécessaire d'améliorer leur coordination la bonne coordination des acteurs et des outils au niveau local doit constituer une priorité l'efficacité de l'ensemble des outils et instruments de prévention des incendies repose en réalité sur une animation cohérente dans les territoires impliquant que l'expertise propres de chacun des acteurs soient valorisés. Telle est l'objet de cet amendement qui concourt à une meilleure préparation de crise ainsi qu'à la planification des moyens des. Monsieur le rapporteur. Merci pour ces deux amendements identiques, le 11 rectifié terre et le 99. Une carte d'aléa a vocation à informer les élus locaux du risque incendie sur un territoire donné. Il s'agit d'un diagnostic objectif du risque. Par conséquent, on voit mal comment une telle carte pourrait être mise en cohérence pardon avec le périmètre des obligations légales de débroussaillement qui sont des mesures de prévention a posée par le code forestier, nous risquons ici d'affaiblir un outil qui sera mis à disposition des élus locaux. Je suis certain que Solène. Cela n'est pas l'intention des auteurs de ces amendements et donc il vous est demandé un retrait ou à défaut un avis défavorable pour ces deux amendements. La ministre. Merci madame la présidente. Monsieur le sénateur Burgos a fait votre avance votre amendement vise à ce que la carte caractérisant le danger de feux de forêt sont cohérentes avec les périmètres soumis. À obligation légale de débroussaillement et qu'elles soient soumises à concertation avec les services départementaux d'incendie et de secours. Le gouvernement partage votre objectif de cohérence et de concertation. C'est dans ce même esprit de prise en compte des enjeux de terrain et de simplification des outils existants que le gouvernement a souhaité préciser par voie d'amendement, le dispositif prévu aux articles 12 et 13 qui ressort des travaux de la commission. Nous vous demandons, comme monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement, je vous remercie. Monsieur quoi. Oui à après les explications de monsieur le rapporteur et de Madame le Ministre je vais retrouver empreint de sagesse. Donc je retire l'amendement. Madame var alias. Qu'en est-il du vôtre. Madame la Ministre m'aurait dit la même chose qu'à monsieur Burgot a puisqu'elle ne m'a pas répondu. Madame la sénatrice var. Je vous dit exactement la même chose effectivement et je vous prie de m'excuser. Merci. Je me vois l'article 13 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 50 Monsieur de Nicolas

Que nous prévoyons à l'article 14 de la proposition de loi porte sur les caractéristiques des constructions même il s'agit par exemple d'intégrer le risque incendie dans le choix des matériaux, la distance d'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de construction par rapport à une parcelle forestière n'a donc peu de Liens avec l'objet principal de cet article 14. Je note de même au demeurant que les élus locaux peuvent déjà sur le fondement de leurs documents d'urbanisme. Interdire les constructions à proximité immédiate des forêts comme le souhaite cet amendement. S'agit donc d'une demande de retrait ou à défaut on chers collègues un avis défavorable. Même avis Madame la Ministre même avis madame la présidente. Pardon. Je me vois l'article 14 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté, le 129 Madame de Marco. Merci la. Présidente du défrichement faut rester lié à l'installation de centrales photovoltaïques sont de plus en plus nombreux, notamment dans le massif landais ou plusieurs milliers d'hectares sont concernés. Après les violents incendies de cet été, de nombreuses propriétaires forestiers sont également démarché par les sociétés qui chassent installer des fermes photovoltaïques sur les parcelles brûlées. Les installations photovoltaïques en zone forestière sont des points sensibles et peuvent s'avérer problématique dans des espaces soumis à un risque de feux de forêt importants. Après de nombreuses questions restent sans réponse. Nous devons rester vigilants. Le rapport que nous doucement donc permettra d'éclairer la situation et de de légiférer en connaissance de cause. Nous avions d'ores et déjà demandé ce rapport lors de l'examen de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Le rapporteur Didier Mandelli nous avait conseillé d'attendre la proposition de loi sur le risque incendie pour aborder ce sujet, aujourd'hui nous y sommes et nous espérons que ce sujet sera pleinement pris en compte. Qu'est l'avis de du rapporteur. Merci madame la présidente. Il s'agit d'une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable sur cette demande de rapport.

qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois l'article 14 bis qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 15, le président Longeau vous avez la parole mais. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues je je tenais à cet article, à prendre la parole. Qu'est-ce qu'un instant. Pour insister sur un le rôle fondamental du débroussaillement d'ailleurs ça a été beaucoup évoqué lors de la discussion générale dans les stratégies de prévention des incendies. j'en profite pour insister devant vous sur le rôle très important que pourrait jouer les personnes inscrites dans un, dans le cadre d'un contrat de réinsertion professionnelle dans ses missions débroussaillement en collaboration bien entendu avec les services de de l'ONF. On sait que le milieu forestier est appelé à. À manquer de bras. D'ici quelques années et il serait intelligent d'orienter dès à présent des moyens financiers qui permettrait de créer de tels contrats pour les personnes en changement de trajectoire professionnelle désireuses de se former à la gestion forestière. On peut encore imaginer que les jeunes inscrits au CNU puisse lors de la 2ème phase obligatoire dites de mission d'intérêt général participer à ces travaux, travaux de sécurisation d'une valeur inestimable pour la préservation de nos forêts françaises. Cela serait complètement en phase avec la philosophie des missions d'intérêt général du SNU et permettrait de sécuriser en urgence de la période estivale des parcelles particulièrement à risque, ces contrats d'insertion ce CNU sont sont vraiment important parce que quand on a nos forêts qui déjà sont beaucoup attaqué par les scolytes et que demain il va falloir mettre beaucoup d'argent pour replanter et si ces replantations sont victimes d'incendies. Donc je pense que c'est une quelque chose Madame la Ministre sur lequel il faut réfléchir et que nous puissions, ensemble, avancer sur ce sujet, je vous remercie. Madame la Ministre, l'amendement 104. Merci madame la présidente. Donc on est sur l'article 15 l'amendement CIV. L'article 15 vise à mieux intégrer dans les documents de planifications et dans les documents Cadre de gestion forestière, de même que dans les PSG des orientations spécifiques aux risques d'incendie. Le gouvernement partage cet objectif afin de préparer au mieux nos forêts face à ce risque qui ne va aller qu'en augmentant. Si l'on se réfère aux dernières projections climatiques cependant certains alinéa de l'article 15 doivent être modifier l'alinéa 3 et La Linea 14 ou supprimer l'alinéa IV à 10 pour prendre en compte les spécificités de chaque document au niveau du Pr FB. Trois ce document n'a pas vocation à établir des prescriptions techniques qui sont du ressort des draps, des DRA TSR. sert GS mais à recenser les enjeux en les croisant au niveau du SR GS. C'est donc une suppression son contenu relève du niveau réglementaire afin de lui permettre d'être ajustés en fonction des différents enjeux forestiers au niveau du PSG. Ce n'est pas le propriétaire qui lui est doté d'un PSG qui doit réaliser travaux de débroussaillement mais le cas échéant, c'est le propriétaire d'une construction voisine. Je vous remercie. et parfois j'encourage. De Nicolas défendu aussi merci. Donc quel est l'avis de la rapporteure. Sur ces trois amendements, merci. Si madame madame la présidente, madame la ministre. Alors sur le quête du gouvernement. Nous y sommes. Opposés puisqu'il nous semble effectivement tout à fait cohérent Madame la Ministre de faire figurer les grands dans les grandes lignes du contenu des des schémas régionaux de Sylvie de de gestion sylvicole dans la loi, notamment en matière de DFCI puisque le contenu des plans Sam de gestion auquel et SRG s'impose figure lui aussi déjà dans la loi. Nous sommes toutefois attaché. À ce que ce passage du réglementaire ou législatif se fassent à droit constant, en y ajoutant uniquement la composante DFCI. Sur le 12 de monsieur Bourgois, il est. Déjà satisfait puisqu'il aborde les sujets de biodiversité qui sont déjà bien présent dans l'est est-ce RJS et enfin celui de monsieur de Nicolas il est dit de Nicolas il est difficile à appliquer. Mon cher collègue, puisqu'il n'existe pas de définition juridique de la libre évolution dans le code forestier et que par ailleurs il impliquerait que finalement toutes les parcelles privées non géré aujourd'hui tomberait sous le coup de cette disposition. Donc c'est une demande de retrait pour les trois amendements sinon un avis défavorable. Bien j'imagine que Madame la Ministre ne retire pas son amendement.

le le 12 et retirer m'a dit, monsieur, bonsoir. Monsieur Nicolas aussi donc il n'y a plus que l'amendement du gouvernement à mettre aux voix qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons au 117 Madame de Marco. Madame la présidente, conformément aux recommandations de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Cet amendement clarifie et renforce l'ambition portée par l'article 15. Pour prévenir et lutter contre une intensification et l'extension du risque d'incendie. Il est nécessaire de favoriser les pratiques civils. Qui améliore la résilience de nos forêts. Il serait dommageable d'encourager à une simple compatibilité entre sylviculture et résilience ainsi cet amendement propose une réécriture plus ambitieuse qui intègre également la notion de changement climatique alors que le dérèglement du climat accroît la vulnérabilité de nos fourrer. Il est nécessaire de l'évoquer dans cet alinéa. Sécheresse maladies ou tempête autant de risques donc la fréquence et l'intensité ne cesseront d'augmenter avec la hausse des températures. En cohérence avec la présente, proposition de loi, il s'agit de réaffirmer l'importance de l'adaptation des forêts au changement climatique.

monsieur, bonsoir. Oui merci madame la présidente. Le schéma régional de gestion sylvicole mériterait d'être transmis au SDIS pour une information à partager visant à une meilleure préparation de crise ainsi qu'à la planification des moyens à déployer, telle est l'objet de cet amendement. Sur. Quel est votre avis madame la rapporteure. Alors je pense que votre en fait votre demande à la satisfaite, mon cher collègue, puisque le SRG s'il est disponible sous forme PDF donc votre amendement reviendrait inscrire dans la loi que le CRPF doit envoyer ce document par courriel. Donc c'est plutôt une demande de retrait un avis défavorable. Comme je suis satisfait. Madame la présidente, je retire madame Manama. Je vous remercie. Deux amendements identiques, le 95. Monsieur gay. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, nous proposons de faire apparaître de façon plus explicite dans les plans somme de gestion. La présence d'éléments indispensables au maintien de la biodiversité, ainsi que les mesures visant à leur préservation en cohérence avec l'action de 3 points de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique, du ministère de l'agriculture et l'alimentation. En favorisant le maintien de la biodiversité, l'adaptation des forêts au changement climatique. Ces éléments participent à la prévention à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Les zones humides, tout comme les gros bois morts au sol permet de conserver l'humidité dans la forêt. De même, plusieurs études ont souligné la plus grande résilience des Grosbois aux incendies. Je vous remercie. je complète pour préserver les éléments indispensables aux écosystèmes forestiers. Il est nécessaire de les identifier clairement leur mention dans les plans simples de gestion permettra de guider les propriétaires et les forestiers dans leurs actions de préservation de la biodiversité. Il s'agit de donner un outil supplémentaire aux acteurs de la. Et de la lutte contre le risque incendie. mes chers collègues, en fait ces amendements sont également déjà satisfait puisque les plans de gestion sont soumis à conformité avec Les SRG S qui eux-mêmes laisse une large place à la biodiversité. Sur les mares forestières les bois mort les îlots de naissance donc ce sera plutôt une demande de retrait ou sinon un avis défavorable. Madame la Ministre même avis même avis madame la présidente. Je vais donc mettre aux voix je mets aux voix ces amendements identiques et pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés je me voir l'article 15 qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté après l'article 15, un amendement 44 monsieur de Nicolas Oui madame la présidente, merci. Il est important que l'ensemble des documents de gestion applicable à la forêt privée, quel qu'il soit intègre cette partie relative aux enjeux défense des forêts des forêts qu'on les incendies. Or l'article fait apparaître les orientations spécifiques au risque incendie dans le plan simple de gestion et le présent amendement vise à les inclure dans les autres documents de gestion que sont le règlement type de gestion et le code de bonnes pratiques sylvicoles de cette manière, l'ensemble des documents, gestion applicable à la forêt privée sont visés tels que cela est prévu par l'exposé des motifs dans la présentation de l'article 15. quel est l'avis de la commission. Selon Madame la Rap un avis favorable puisque la l'amendement notre collègue vient utilement compléter notre rédaction. Madame la Ministre, avis favorable du gouvernement. Vous voyez Monsieur de Nikolaï. Je le mets donc aux voix double avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Ensuite, nous avons l'amendement 36, qui le défend Madame Lazard a trouvé moi même. Si depuis plusieurs années le seuil d'acheter le seuil d'assujettissement au plan Simple de gestion ne cesse de se complexifier, d'évoluer, ce qui pose plusieurs difficultés. En 1er lieu les Centres régionaux de la propriété forestière n'ont toujours pas terminé les appels auprès des différents propriétaires forestiers pour les informer qui sont dans l'obligation de détenir un plan simple de gestion depuis la réforme résultant de la loi de modernisation agricole 2010 et le décret du 25 mai 2011. Ensuite les propriétaires forestiers commencent à manquer de visibilité avec l'ensemble des refontes concernant les documents de gestion durable. Les codes de bonnes pratiques sylvicoles devons obligatoirement prévoit un programme de coupes et de travaux depuis la loi du 25 août 2021. août 2021. Tout en reconnaissant l'intérêt des documents de gestion durable leur propre leur portée effective en matière de prévention incendie reste insuffisante. Par conséquent, cet amendement propose de supprimer l'article 16. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Alors ce sera un avis défavorable puisque la la commission c'est la c'est prolonger prononcée favorablement pour un, un abaissement du seuil des plans de gestion à à 20. Attends je rappelle d'ailleurs comme l'a évoqué, Madame la Ministre tout à l'heure que c'était une des conclusions phare des assises de la forêt et du bois partagée par l'ensemble des professionnels cette ce rabaissement du du du seuil des plans de gestion permettra à 20.000 propriétaires de rentrer dans une démarche de documents de gestion durable et donc de 500 à 500.000 hectares d'être suivis régulièrement et depuis de pouvoir être pleinement intégré à la logique DFCI. Donc c'est vraiment une demande de retrait ma chère collègue ou sinon un avis défavorable.

Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté à l'article 17 l'amendement huit Madame de Marco. Merci à travers cet amendement, nous souhaitons donner plus de force à la traduction de la recommandation numéro 38 du rapport d'information de la mission conjointe de contrôle. Pour mieux distinguer l'essentiel de l'accessoire, il est proposé que la puissance publique. Autrement dit, le Centre régional de la propriété forestière hiérarchise les enjeux des modèles de plans de gestion en insistant sur leur orientation en matière de protection des forêts contre l'incendie. Au lieu de simplement invité des propriétaires et gestionnaires à le faire. La montée en puissance des documents de gestion durable doit effectivement s'accompagner d'une mise à jour sur le contenu les priorités du plan enceinte de gestion doivent être davantage orientée sur la protection et la défense de la forêt contre les incendies. Cet amendement vise ainsi à faire de la lutte contre le risque incendie, une des priorités de la gestion forestière. Merci que l'avis de la commission, madame la rapporteure. Alors ce sera un avis plutôt défavorable, parce que le le rôle du CRPF ni de pas de 2 hiérarchiser mais bien de vérifier la conformité et l'application notamment une fois encore des principes inscrits dans le schéma régional de gestion sylvicole et s'il estime que les principes hein. Tant sur ce territoire et inscrit au schéma d'de j'régional de gestion sylvicole ne sont pas. Ne sont pas suivis il pourra à ce moment-là ne pas donner l'agrément, donc c'est plutôt une demande de retrait sinon un avis défavorable, parce qu'en fait ce contrôle sera fait a posteriori par le CRPF. Madame la Ministre. Merci madame la présidente chez madame la sénatrice de Marco. Un complément. Des propos de Madame la rapporteure et avec un avis défavorable aussi mais quelques explications. L'objet. Fixé au Centre national de la propriété forestière depuis 2012 par sa tutelle et de veiller à ce que tous les centres régionaux utilisent le même modèle de PSG, de manière à homogénéiser les outils et les pratiques. Cela est d'autant plus important aujourd'hui dans le cadre de la dématérialisation des PSG qui nécessite un modèle unique la hiérarchisation des enjeux doit bien être adaptées à chaque situation forestière et c'est donc bien au propriétaire aider éventuellement d'un expert de procéder à cette hiérarchisation, la protection des forêts contre l'incendie était évidemment le sujet du jour mais nous nous devons de veiller à l'équilibre entre les différents enjeux et je ne peux pas soutenir une inclusion spécifique au niveau des enjeux du PSG ouvrir à un caractère obligatoire de l'orientation même pour un motif tels que la prévention des incendies, nous semble par ailleurs une atteinte disproportionnée au droit de la propriété, garanti par notre Constitution. Aussi, le Gouvernement émet un avis. on voit maintenant pendant le 85 de Monsieur Gillet. Merci madame la présidente madame administre madame la rapporteure. Cet amendement nous tient à coeur qu'elle révise à prendre en compte le phénomène d'illectronisme encore très présent en France. Nous sommes tous conscients que l'avenir passe davantage par la dématérialisation pour faciliter l'accès, information et ça présente un certain nombre d'avantages environnementaux. Donc il y a pas de de questions par rapport à ça pouvons pouvons tous ceux constatés dans nos territoires que l'accès Internet reste très inégale et que certains publics faute d'accompagnement non pas nécessairement franchi le pas du numérique. Je vous rappelle qu'à peu près 25% de personnes qui sont en situation de décrochage, en conséquence nous souhaitons préciser la rédaction d'articles 17 qui prévoit que le CRPF met à disposition des propriétaires sous forme dématérialisée des modèles de plan simple de gestion pour les accompagner au mieux et leur permettent de hiérarchiser les enjeux. Nous souhaitons donc maintenir ce principe général, mais prévoir en cas d'impossibilité pour un particulier, d'avoir accès de façon dématérialisée au document la possibilité de se rendre en maison de service au public ou bien en sous-préfecture pour se les procurer en format physique. Il s'agit là de n'exclure personne en termes d'accessibilité. Alors en commission, nous avions valider votre amendement, mon cher collègue. S'il y avait un certain nombre de de de rectification et je ne je je vous ne les avait pas évoqué. Qui était que nous laissions en fait. Alors s'agissant uniquement des propriétaires particuliers puisqu'en fait pour tous les autres propriétaires ils ont recours à des gestionnaires, voire à des coopératives donc ils peuvent tout à fait remettre les documents sous forme dématérialisée, mais pour répondre à votre demande légitime, nous vous proposions un dispositif spécifique pour les propriétaires particuliers avec une remise au CRPF. Juge et avec un report de l'option dématérialisé jusqu'en 2030. Donc si vous êtes d'accord sur cette rédaction c'est un avis favorable. Je vous remercie madame la rapporteure effectivement je suis favorable. Document, on était pas mis à jour. Je vous remercie. Oui mais on aurait besoin qu'elle soit. C'est. C'est monter.

Donc seul le Centre régional de la propriété foncière est habilité le plan Simple de gestion la télé-déclaration de ces plans est un levier fort pour encourager la gestion durable de la forêt privée, laquelle doit contribuer à réduire le risque incendie dans les massifs concernés dès lors il n'apparaît pas opportun de prévoir la possibilité d'une remise de ces plans sous forme papier aux maisons de service au public et aux sous-, préfectures, des points d'accès ou d'aide au numérique dans tous les territoires comme les maisons de service public peuvent par contre être des lieux où les personnes éloignées du numérique peuvent remplir leurs obligations de plus les experts forestiers ou coopératif peuvent également télétransmettre au nom du propriétaire, donc nous émettons un avis de sagesse.

cette rédaction convient. À Monsieur Gillet et ses co-rédacteur Madame la Ministre vous aviez émis un avis de sagesse. J'imagine que ça ne change rien. Je vais le mettre. Au revoir. Donc. C'est un amendement maintenant qui coproduit par la commission et Monsieur Gillet, avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 17 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Madame de Marco le 119. Merci. Nous saluons la consécration du principe des visites à mi-parcours déjà mises en oeuvre dans certains territoires dans la limite des moyens disponibles et la généralisation du droit à une telle visite. Il s'agit ici d'apporter un complément dans cette fonction de conseil auprès des propriétaires forestiers. Nous souhaitons que la visite et le bilan à mi-parcours de l'exécution du plan de gestion par un technicien forestier encourage les méthodes sylviculture qui s'appuie sur les fonctionnalités des écosystèmes. Pour que cette fonction du Conseil prenne tout son sens au regard du but poursuivi par cette proposition de loi, il semble nécessaire de mentionner ses objectifs à 100, puis en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature les fourrer plus résilientes face à de multiples Alder aléas sont en meilleure santé sont dans moins combustible. De plus, des pratiques civils colle plus durable devrait permettre de pouvoir réconcilier les enjeux de lutte contre les risques d'incendie et de préservation de la biodiversité. Il s'agit aussi par cet amendement de garantir que la valorisation économique Dubois et de la biomasse biomasse ne soit pas la seule boussole pour guider propriétaires forestiers dans les dicussions du du document gestion durable. Nous voyons ici en creux une vision productiviste de la forêt qui ne pas souhaitable. Enfin, cet amendement permet de concilier concrètement la lutte contre les incendies et la protection de la nature et de la biodiversité. Ce sera une demande de retrait un avis défavorable pour les mêmes raisons que celle qui a déjà été évoquée. Chers collègues, c'est que c'est l'essence même je dirais. Du CRPF que de prodiguer des conseils qui tiennent compte des fonctionnalités des écosystèmes de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique et c'est tout l'intérêt de cette visite à mi-parcours aujourd'hui justement pour pour venir ajuster un petit peu les préconisations auprès des des propriétaires donc c'est je dirais que votre amendement et en fait déjà satisfait donc c'est plutôt une demande de retrait ou un avis défavorable.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Mais le va Madame de Marco. L'alinéa 5 de l'article 18 propose de renforcer les aides publiques aux associations syndicales de gestion forestière. Dans le cas de l'application de leur plan Simple de gestion afin de rester en cohérence avec l'objectif de cette proposition de loi. Nous souhaitons limiter cette majoration d'aide publique aux actions de défense des forêts contre les incendies. Toutes les actions prévues par le sang plein plan simple gestion ne sont pas profitables à la lutte contre le risque incendie, l'argent public doit soutenir des pratiques action civile cols les plus vertueuses. Si, quel est votre avis madame la rapporteure. Alors ce sera idem hein. Une demande de retrait ou un avis défavorable puisque cette proposition reviendrait pas finalement à restreindre en pratique le le financement de la valorisation économique de la forêt qui je le rappelle, fait fait partie de la bonne gestion durable de la multiplication fonctionnalités des forêts et elle contribue donc plus ou moins directement mais en tout cas à la bonne gestion et donc à la défense des forêts contre les incendies. Donc c'est plutôt un avis défavorable demande de retrait le ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice de marque. Pour la mutualisation coffre l'existence du Nasa présente un réel effet de levier pour augmenter le taux de couverture des forêts privées par un document de gestion durable. Un tiers seulement des forêts privées ont aujourd'hui un document de gestion durable et la limitation de la bonification proposée par l'article aux seules actions DFCI paraît logique, même si sa mise en oeuvre. On n'est pas forcément aisée. Dès lors que la gestion forestière forme tout répondant des différents enjeux l'de la mention n'apparaît donc pas du tout utile. Donc, avis défavorable comme la commission. Je mais voit double avis défavorable qui pour. Qui est contre qui s'abstient pas adopté de 68 madame arriver. c'est un amendement de d'appel et au terme de mon explication je le retirerai puisqu'il a déjà un, un avis négatif. C'est une demande de rapport pourquoi parce que l'article 18 prévoit dans le cadre des PSG un accompagnement des propriétaires forestiers par la visite d'un technicien forestier du CNPF à mi-parcours, cette visite doit faire l'objet d'un bilan dans le but d'encourager les méthodes de sylviculture durable. Nous sommes favorables au dispositif tels qu'il a été prévu. Pourtant, nous voulions attirer l'attention du gouvernement sur les moyens humains du CNPF et son adéquation avec l'ensemble de leurs missions qui sont croissantes. Il faut rappeler que 75% de la forêt française et privés. Elle représente ainsi 23% du territoire, 12 millions d'hectares et cette forêt privée très morcelé compte 3 5 millions de propriétaires avec en moyenne 3 4 hectares de surface par propriétaire avec 350 équivalents temps plein une vino les moyens humains du CNPF semble ah déjà assez contraint et donc si on leur donne des missions supplémentaires, ça risque de poser problème. Le CNPF a été épargné en 2023 grâce à la mobilisation du Sénat. Lors de l'examen du PLF, et nous saluons ici le travail des sénateurs en particulier de notre collègue Jean-Claude Tissot co-, rapporteur pour avis du budget agricole, donc l'objectif de cet, de cet amendement. C'est demandé un rapport pour avoir vraiment les éléments mis sur la table par le gouvernement en terme de moyens mais je le retire puisqu'il s'agit d'un rapport et qui leur il aura bien entendu un avis négatif à la fois de la commission, ça je le sais déjà et du gouvernement. Merci. Juste insister parce que je crois que ma chère collègue. Vous avez raison d'insister sur les besoins de financement dont nous reparlerons lors du prochain PLF mais derrière cette PPL il y a effectivement des besoins d'abondement au CNPF allait à l'ONF et j'ai l'ensemble des acteurs forestier néanmoins peut-être pour vous, vous avez une information, je pense qu'on a sur le fond, pas forcément besoin d'un rapport. que s'agissant du CNPF, on compte des demi-journées de de consultation par le nombre de PSG donc on arrive à quantifier les besoins sans forcément qu'il y ait un rapport en tout cas, vous avez raison de soulever ce, ce sujet majeur. Madame la Ministre vous souhaitez. Oui, mais vous pourriez néanmoins avoir.

Bien. L'article 18 je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté l'amendement 147 Madame Loisy madame la rapporteure. Il s'agit d'un complément. Donc à à l'article 19 l'ajout des entreprises de travaux forestiers dans la liste des personnes avec lequel le réseau de référents DFCI du CNPF devra se concerter. Madame la Ministre, quel est votre avis. Sagesse. Je mets aux voix cet amendement de la rapporteure avec sagesse du gouvernement qui est. Pour qui est contre qui s'abstient. Il était adopté. Le quatre. Madame la Sarah c'est vous qui le défendait. Vous en êtes la troisième non oui non pour Union. Mais même leur toutes nos excuses. Merci. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Cet amendement a pour objet d'intégrer les exploitants forestiers à la gouvernance de la prévention des incendies en effet les rapporteurs ont introduit un amendement en commission qui prévoit que le Centre national de la propriété forestière CNPF puisse mener des concertations avec les parties prenantes, telles que les associations syndicales mentionnés à l'article L 132 tiré de du code forestier, les services départementaux d'incendie et de secours. Les gestionnaires et propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l'Office national des forêts. Pour compléter cette liste. Je propose d'y intégrer les professionnels de la forêt privée qui ont un rôle clé dans le dispositif de lutte contre les incendies et qui ont largement oeuvré lors des feux de forêt or nomme hors norme en Gironde et dans les Landes durant l'été dernier 2022 ce sont des acteurs essentiels puisque le cadastre. Recense 3 8 millions de propriétaires forestiers qui possède près de 76% de la surface forestière privée. Ils ont une connaissance précise des parcelles et leur présence quotidienne sur le terrain permet d'identifier les risques de départs d'incendie. Ils peuvent également guidé les pompiers dans leur mission. Et enfin, il possède le matériel nécessaire pour intervenir en cas d'urgence. Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable de les associer en amont à la prévention et à la lutte contre le risque incendie. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure. Alors, mes chers collègues, nous avons je pense largement répondu à votre demande par l'amendement qui vient d'être voté et qui intègre donc les entrepreneurs de travaux forestiers, les entrepreneurs de travaux forestiers. Ce sont les entreprises qui font des prestations de service pour les propriétaires qui sont donc au quotidien dans les forêts sur les parcelles et qui font de l'entretien, les exploitants, les entreprises qui sont uniquement que je porte dans forestier, beaucoup d'exploitants sont en fait entrepreneurs parce qu'ils font des travaux et ils font du négoce, les exploitants forestiers quand ils sont uniquement exploitant forestier, ce sont des gens qui font du négoce, donc ils ne sont pas au quotidien dans les forêts et ils ne connaissent pas particulièrement les massifs. Ils ne seront pas forcément en contact avec les propriétaires. Donc ce sera plutôt une demande de retrait sinon un avis défavorable. Ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Votre amendement propose ajouter parmi ces acteurs les exploitants forestiers. Ses exploitants forestiers peuvent en effet à la demande des propriétaires forestiers assurer une partie des travaux forestiers pourraient ainsi être utile qu'ils puissent échanger avec le CNPF, et par exemple, identifier les parcelles présentant une vulnérabilité aux incendies afin qu'une action d'information et de sensibilisation soit faite auprès des propriétaires des dit. Parcelles toutefois semble-t-il de rappeler que l'organisation de la politique de défense des forêts contre les incendies ne relève pas du niveau législatif nous émettons un avis de sagesse.

Ils sont à intégrer dans ce dans dans ses. Ils sont pas référent, il devrait être partie prenante. Merci. Je mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour.

Lors de ces travaux. La mission flash incendie de feux de forêt, l'association de des départements de France, a insisté sur un meilleur partage des informations et à l'émergence d'une culture du retour d'expérience afin de confronter les plans existants à la réalité pratique en ce sens bien sûr le retour d'expérience et. Prioritairement à faire émerger des pistes de progrès utile localement et dans un second temps, à faire l'objet d'une analyse au sein de l'administration centrale afin de capitaliser sur les bonnes pratiques, d'une part et de prendre en compte les problématiques récurrentes. D'autre part le retour d'expérience, bien sûr il continue il contribue à optimiser sur le plan humain organisationnel et technique. Le fonctionnement des organisations qui concourent aux missions de prévention et de lutte contre les incendies. C'est la raison pour laquelle il est proposé par cet amendement que le coordinateur au niveau central chargé de la mutualisation des retours d'expériences entre territoires transmettre ce document à l'ensemble des départements pour un échange de bonnes pratiques entre eux. Donc je me suis. Des. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements.

Plus tôt au Conseil gêné départementaux et pas directement au SDIS en fait qui sont quelque part les bras opérationnel des départements en matière de sécurité des biens et et des personnes. Donc ce sera plutôt une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable, sachant que bien évidemment ces documents peuvent être transmis une fois encore, sans pour autant qu'il soit inscrit dans la loi. Et sur le. Sur le. 14 madame la. Rapporteure.

Qui contre. Qui s'abstient. Il n'est pas l'adopter. Le 14 et retirer et je mets donc aux voix l'article 19 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté Maintenant le l'amendement 121 madame de Marco. Merci madame la présidente. Le crédit d'impôt au titre des investissements forestiers conditionnée à l'application d'un plan de gestion. Si aucun plan simple digestion ni gris au moment de l'acquisition du terrain. Le propriétaire a un délai de 3 ans pour le faire agréer. Cet amendement propose de réduire le délai prévu en passant de 3 à 2 ans. Le plan celle de gestion et garant d'une gestion durable de la forêt. Il peut également jouer un rôle important dans la prévention et la lutte contre le risque incendie, il est nécessaire que les forêts concernées par ce crédit d'impôt s'inscrivent au plus vite dans une démarche de durabilité de résilience un délai de 2 ans pour faire agréer un plan ça de gestion semble suffisant. je ne suis pas certaine ma chère collègue que ce soit très opportun de réduire ce délai puisque l'article 16. Nous venons de créer quelque part un appel d'air avec 25.000 nouveaux plans. plans. De gestion qui vont arriver sur le bureau. En tout cas des des des différents CRPF. Et sachant que pour faire un plan de gestion, ça prend du temps, il faut trouver un gestionnaire. Il faut que le gestionnaire viennent sur les parcelles. Ça peut prendre de longs mois, voire plus d'un an pour faire un plan de gestion d'une grande forêt. sans aucun problème. Donc je je vous poserais plutôt de le retirer, parce que je pense que trois ans ne seront pas superflus dans le contexte Post-article 16 surtout. Madame administre. Merci madame la. Président en complément, rappeler que la loi de finances pour 2023 vient juste de proroger simplifier et renforcer le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier madame la sénatrice de Marco. Le gouvernement n'entend pas revenir sur les paramètres de ce dispositif pour laisser aux acteurs le temps de s'approprier cette réforme toute récente donc dans ces conditions nous. Nous demandons de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous vous mettons et mettrons un avis défavorable. Monsieur Gillet pour une explication de vote. Merci madame la présidente, très rapidement. Oui mais là on est bien adossée à un crédit d'impôt donc un plan sorte de gestion participe effectivement d'une lutte intéressante. Au niveau des incendies. Donc le fait d'y adosser un crédit d'impôt, il est quand même logique, à un moment donné, on essaie de se mettre en conformité le plus rapidement possible de les deux ans est quand même pas incontournable. Donc je vais mettre aux voix cet amendement. Qui a reçu double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 134 Madame de Marco. Merci. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de l'article 35 de la proposition de loi qui conditionne les aides publiques, un mélange d'essence en forêt. En effet, cet article pour nous va dans le bon sens, celui de conditionner les aides publiques à la mise en oeuvre une gestion des forêts plus multi-fonctionnel et qui favorisent la résilience. Si l'article 35 est un 1er pas nous souhaitons notamment sur le crédit d'impôt défi acquisitions et travaux, aller plus loin dans la conditionnalité pour Fabrice. Vous visez la résilience des forêts. Ainsi, nous proposons que soit mise en place pour ce crédit d'impôt une conditionnalité environnementale est lié au risque incendie qui soit, et notamment sur la gestion civile avec un véritable mélange d'essence mais aussi l'absence de coupe rase hors motifs sanitaires. Les pratiques civils colle plus proche de la nature permettent, en plus de présenter un intérêt environnemental une meilleure résilience des forêts à différents aléas tempête risque sanitaire, changement climatique et présenter des atouts dans la gestion du risque incendie. Ainsi, par une autre conjointe, le comité français de l'UICN et la Société botanique de France estime que la pratique des coupes rases et les monocultures en plus d'avoir des effets néfastes sur la biodiversité ne sont pas un atout pour la gestion du risque incendie alors que les pratiques civils colle plus durable et notamment basé sur le mélange d'essence de la sylviculture a couvert continue devrait permettent de réconcilier ces enjeux c'est assez assez. Dans cet esprit que nous proposons de conditionner ce crédit d'impôt.

Il nous semble qu'il est important de préserver la diversité des modes de gestion en adéquation aussi avec des réalités des territoires qui parfois justifie des modes de gestion diversifiée. Je vous je souligne que par ailleurs nous avons refusé d'un d'interdire la libre évolution. Donc nous ne sommes pas dans une stratégie nous interdisons telle ou telle pratique et nous laissons aux acteurs de terrain. Le choix de l'opportunité des des bonnes pratiques. Je souligne également que votre amendement est tout de même partiellement satisfait puisque à l'article 35. Nous verrons tout à l'heure nous introduisions des conditions globales sur des principes de diversification des essences. y compris pour le crédit d'impôt et que notre rédaction de commission que nous avons précisé en séance clarifie que la régénération naturelle donne bien droit. Ah l'accès au à la défiscalisation dispositif défi donc ce sera plutôt une demande de retrait sinon un avis défavorable. merci Madame la Ministre même avis madame la présidente. Je mais aux voit double avis défavorable qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 148 madame la rapporteure. il s'agit d'un d'un complément. De l'éligibilité au sens large des dépenses de travaux forestiers tout en maintenant la mention explicite des travaux favorisant la régénération naturelle et les regards ni de plantations. Madame la Ministre, quel est votre avis. Malheureusement, nous demandons à madame la sénatrice loisir de bien vouloir retirer. Cet amendement pour les mêmes raisons que celles que j'ai. Indiqué tout à l'heure, l'article 10 de la loi de finances pour 2023 prorogé simplifier significativement renforcer le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier. Donc nous souhaitons, nous ne souhaitons pas revenir sur les paramètres de ce dispositif, parce qu'il est extrêmement récent pour laisser aux acteurs le temps de s'approprier cette réforme ambitieuse. L'entrée en vigueur est extrêmement récente. Donc, nous vous demandons de bien vouloir le retirer et à défaut, nous voterons défavorable. Et donc mettre aux voix cet amendement de la rapporteure avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté l'article 20 qui est pour. Ce qui est contre qui s'abstient il est adopté après l'article 20 l'amendement 22, madame la présidente Delattre. merci madame la présidente, mes chers collègues, à ce jour, seuls les sylviculteurs du Sud-Ouest sont assujetties depuis 1945 à une taxe de défense des forêts contre les incendies. Pour la mise en défense de la forêt. Cette taxe est censé dégager des marges de manoeuvre financières pour les protéger d'un risque pour lesquels ils ne sont pas fautifs. En effet, les départs de feu sont majoritairement de nature humaine et le plus souvent exogène au milieu forestier et donc ils subissent et supporte des feux. D'origine donc comme je viens de le dire exogènes dans un souci d'équité, de bon sens. Il apparaît opportun qu'une défiscalisation de la taxe de DFCI soient mises en place, loin d'être une niche fiscale déguisée, elle permettra aux sylviculteurs d'investir davantage dans la protection et l'entretien de leurs forêts. Je vous remercie. merci. Quel est l'avis de la commission. soit intégralement donc je suppose. Par le contribuable. Donc ce sera. Une défiscalisation à 100% serait un autre sens excessive et. Et et difficilement justifiables. Donc ce sera plutôt un avis défavorable. Madame la ministre, même. Même avis madame la présidente. Je mets aux voix, madame la présidente. Double avis défavorable. Qui est pour. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté après l'article 20. Nous avons 2 amendements en discussion commune le 88 Madame Breillat. de loi de finances en en rapport, nous ne cessons de le répéter qu'il est fondamental de préserver les capacités humaines et matérielles de lutte contre les incendies. à cet égard la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie du Sénat du 3 août 2022. Demander de revenir à minima sur la suppression des 500 postes prévus à l'ONF, nous le savons tous. Le rôle de l'ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentielle. Or l'adoption du nouveau contrat État ONF acté la suppression de 500 postes d'ici 2025 alors même que l'organisme est exemple ainsi en dépit de son importance stratégique. L'ONF et pourtant la cible d'une politique d'affaiblissement continu cette perte d'effectifs et d'expertise s'avère dangereuse. Les forestiers sont en première ligne pour alerter les départs de feu les combattre avec des patrouilles prépositionnés. Le département recherche et développement de l'Office national des forêts doit également être renforcée et malgré cela, nous constatons que les décisions de réduction d'effectifs prises vont à l'encontre de toutes les recommandations. Oui, c'est effectivement le mène à mon demain je vais apporter des arguments complémentaires. L'Office national de forêts doit avoir des moyens suffisants pour exercer l'ensemble de ses missions, en particulier en matière de prévention des risques et de constatation des infractions forestière comme la non-, réalisation des obligations de débroussaillement. Il importe de redéployer dans l'ensemble des forêts publiques. Un certain nombre d'agents de surveillance au sein de l'ONF dont les effectifs ont été limités ces dernières années. Les nouveaux défis auxquels est confrontée la filière bois, parmi lesquels des dépérissements et les incendies liés au changement climatique en chambre d'une nouvelle mission confiée à l'ONF. Il s'agit aussi de traduire dans la présente, proposition de loi la recommandation numéro 16 du rapport d'information de la mission de contrôle à l'origine de cette proposition de loi. J'en rappelle ici le contenu. Entrée guillemets revenir sur les 500 suppressions de postes de l'ONF prévue dans le contrat État ONF 2021 2025 pour établir des postes d'agents de protection de la forêt méditerranéenne supprimer ces dernières années et redéployer plus de postes sur expertise DFCI aux régions méditerranéennes, en étant dans le périmètre géographique de la mission d'intérêt général DFCI à l'ensemble du territoire national, je ferme les guillemets cet amendement vise aussi à mettre les moyens de l'ONF, un accord avec ses nouvelles missions. Il précise, il précise que le contrat pluriannuel passé entre l'ONF et l'État détermine les moyens financiers et humains. Par l'État pour l'accomplissement des missions de l'ONF que celle-ci lui soit confiée par la loi ou qu'elles relèvent des missions d'intérêt général confiée par l'État. Je vous remercie de l'avis de la commission sur ces amendements. Alors sur ces deux amendements. La commission partage. La préoccupation de de nos collègues, s'agissant des moyens financiers et humains accordée à à l'ONF. Néanmoins, nous l'avons déjà évoqué en commission, cette proposition de loi n'est pas le le vecteur adéquat, nous aurons à. À à débattre et à défendre ses propositions lors du prochain PLF donc ce sera plutôt une demande de retrait sinon un avis défaveur. La ministre. Demande de retrait sinon défavorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix d'abord l'amendement 88 d'avis défavorable pied pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le trois même vote. Même vote n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 20 bis qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté à l'article 21. Madame la présidente Delattre l'amendement 26. Trois amendements identiques et vous comme c'est vous. Merci madame la présidente, mes chers collègues. Actuellement, le code forestier, prévoit que l'autorité administrative compétente de l'État élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, l'article 21 de la proposition de loi prévoit une déclinaison de ce plan en différents plans de massifs établissant donc pour chaque massifs forestiers homogène. Une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier en commission, le Sénat a modifié cet article. À la suite d'un amendement que j'avais déposé en prévoyant d'inclure les chambres d'agriculture dans la stratégie du collectif concertée établi pour chaque massifs forestiers homogène et je vous en remercie. Je pense que nous pouvons encore ouvrir la liste des organismes participant à élaborer cette stratégie collective concertée en incluant les structures des Zaza DFCI et le regroupement. Je vous remercie. Sagesse je mets donc on voit ces trois amendements identiques, avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement madame la présidente Delattre. Vous êtes vous vous apprêtez à voter avec enthousiasme. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils sont donc adopté. Madame de Marco de 131. Cet amendement a pour but d'associer plus largement le monde agricole, la concertation sur les risques incendie, cela a été dit, il est nécessaire de construire des synergies avec le monde agricole pour lutter plus efficacement contre le risque incendie. Encore une fois, nous pensons que d'autres acteurs agricoles en complément des chambres d'agriculture doivent apporter des éléments intéressants. La concertation. Cet amendement propose donc d'inclure les organisations professionnelles agricoles et notamment les organisations représentant le pastoralisme à la concertation prévue à l'article 21 sur les plans du massif. Nous l'avons dit, la diversité des agricultures et des systèmes agricoles est en effet intéressant à prendre en compte pour la gestion du risque incendie efficace et en particulier le pastoralisme qui permet de concilier production agricole et débroussaillement. Sur de nombreux territoires, les acteurs du système pastoraux participe déjà avec efficacité la lutte contre le risque incendie en partenariat avec l'ONF ou des collectivités. Il est donc légitime de les associer à la concertation et ce d'autant plus qu'ils souffrent d'un manque accru de soutien de politiques publiques, notamment du fait de la déclinaison française de la politique agricole commune. Cette tendance va à rebours de la prise en compte des enjeux de la biodiversité de production. École durable mais aussi de gestion du risque incendie. Ils font donc enrayer comme le propose. Il faut donc Ce sera un avis défavorable, ma chère collègue puisque nous, nous pensons que la représentation la session des Chambres d'agriculture répond déjà à votre demande. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice de marque. En fait, votre amendement propose d'inclure explicitement des représentants des organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des acteurs pastoraux lors de la concertation permettant la déclinaison des pépés FCI en plan massif dans sa rédaction actuelle. L'article 21 ne prévoit pas cette participation qui nous semble tout à fait pertinente. Vu l'importance de l'interface entre les zones agricoles pour ces raisons et comme je l'ai fait pour l'amendement 130 que vous avez déposé à l'article 1er, je donne un avis favorable à votre amendement. Alors je vais donc mettre aux voix cet amendement 131 qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Madame la. Portable. Donc qui est pour. On va compter là. Qui est contre.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté après l'article 21, un amendement 27. Madame. Amendements identiques, et le 27 de la madame la présidente Delattre. Ou le 34 de Madame Lassaad. Oui merci madame la présidente, mes chers collègues. L'objet du présent amendement et de reconnaître légalement l'activité les travaux réalisés par les associations syndicales autorisées les Zaza de défense des forêts contre l'incendie dans les massifs, organisés autour de ces associations. Cet amendement et d'abord l'occasion de saluer l'ensemble des travaux réalisés par ses Zaza qui depuis plus de 50 ans facilitent l'accessibilité des territoires sur lesquels elles interviennent à travers un réseau de voies susceptibles d'être utilisés en intervention dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces chemins piste route forestières sont regroupés sous l'appellation de voix d'intérêt opérationnel aujourd'hui mais ce seul statut ne permet pas de les protéger suffisamment ni matériellement ni juridiquement aussi l'objet de cet amendement et de les reconnaître légalement. Ainsi, d'une part les voix défense des bois et forêts contre l'incendie créée par ces associations bénéficieraient d'un statut de voix spécialisée non ouverte à la circulation générale. D'autre part, il serait interdit aux propriétaires de terrain de modifier librement la continuité des ouvrages Aménagement et travaux de prévention des bois et forêts contre l'incendie. Les modifications ne pourrait résulter que d'une décision de Lhasa je vous remercie. Je rajouterai simplement sur l'amendement identique que. Cette ces dispositions. N'entraînerait aucune dépense additionnelle. Très bien quelle est la position de la commission, madame la rapporteure. que mentionne donc vos amendements et les voix de défense des bois et forêts contre l'incendie, déjà reconnue par le code forestier en son article 134 de dons l'établissement relève de la compétence de l'État, et parce qu'elles sont établies au nom de la puissance publique que les voix DFCI ont déjà le statut de voix spécialisée non ouverte à la Syrie. Population générale conformément donc à l'article 134 tiret 3 du code forestier. Je note par ailleurs que vos amendements sont finalement sur le fond largement satisfait puisque le même code forestier dispose que les voix des filles qui prennent la forme d'une servitude de passage et d'aménagement sont certes établi par l'État mais et que cela peut l'être en fait des associations syndicales donc pour ces raisons, ce sera une demande de retrait sinon un avis défavorable. Ministre même avis. Je mais on voit ces deux amendements identiques, qui ont reçu. Hier. Vous aussi, madame la présidente. Donc ils sont retirés à partir que le 22 madame Jourdain, vous avez la parole. parole. Madame la présidente. Mes chers collègues. Un mot pour réaffirmer l'attachement des communes forestières pour cet article 22. En effet celui-ci institut un droit de préemption pour les communes lorsque sur les parcelles concernées, un, un jeu a été préalablement identifiés comme stratégique au regard au regard de la défense des forêts contre les incendies cet article que constitue un outil indispensable dans la protection de leur territoire et de la population. Nous vous invitons en conséquence en le mettant à le

Des communes disposent également d'un trois de préférence en cas de vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares situés sur leur commune. Par ailleurs le droit de préemption de l'est et le droit de préférence des propriétaires forestiers, voisins sont également applicables en cas de vente de parcelles d'une super d'une superficie inférieure à quatre hectares. L'ajout d'un nouveau droit de préemption au profit des communes basée sur des conditions différentes entraîne une complexité juridique supplémentaire lors des opérations de cession de parcelles boisées de plus ce cumul de droit de priorité entraîne alors un allongement du délai de réalisation des opérations de cession difficilement compréhensible pour les partis à l'acte dès lors que l'opération porte sur une parcelle de faible superficie. Alors c'est un avis défavorable puisque avec ce droit de préemption DFCI, nous répondons à une attente forte. Des élus des communes forestières pour leur permettre de faire valoir donc un droit préemptions dans le cadre de surface et de parcelles qui présenteraient des dangers. DFCI. Dans le cadre, je le rappelle d'un document d'un cadrage PPCI ou. Donc c'est une mesure qui aura un caractère exceptionnel et qui permettra aux communes de ne pas subir et la présence de parcelles dangereuse sur des périmètres identifiés comme étant à risque sur des terrains communaux. Et donc, j'insiste sur le fait que le cadre au Sahara essentiellement celui des pépés fille ou des prix. Il s'agit pas d'un droit de préemptions DFCI ouvert sur tout l'Hexagone, mais uniquement dans le cadre de préconisations d'un d'un document DFCI. DFCI. La ministre même avis. Oui l'idée ça serait plutôt de demander à monsieur Duc de Nicolas il de bien vouloir le retirer au profit de l'amendement suivant de Madame Loisier le 149. Sinon défavorable. Ces 3 dames qui me le demande j'accepte. Très bien. Moi-même je ne dis rien alors ne dites rien non plus. Bien madame. Voyez bien présenter votre amendement 149. Au profit duquel monsieur Nicolas. Théoricien. Alors il s'agit d'un amendement effectivement qui revient sur le droit de préemption DFCI des communes. Et qui en précise les modalités et notamment le fait que ces propriétés seront soumises au régime forestier et administré conformément à celui-ci. Madame la Ministre, j'ai cru comprendre favorable ensemble. Je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 22 qui est pour et contre qui s'abstient il est adopté à l'article 23. Madame de Marco l'amendement 122 merci. Si cet amendement vise à préciser que les mesures de prévention intégrer dans les stratégies locales développement forestier s'appuie en particulier sur les solutions fondées sur la nature ou les fonctionnalités des écosystèmes préserver la ressource en bois des incendies. Il s'agit tout simplement de renforcer l'objectif poursuivi par la petite le 23. Si madame la rapporteure. Quel est votre avis. Sera un avis plus. Défavorable, parce que nous sommes satisfaits madame chers collègues puisque les les missions des stratégies locales de développement forestier sont d'ores et déjà de garantir la satisfaction des demandes environnemental ou social concernant la gestion des forêts des espaces naturels qui leur sont. Connexes, donc ce sera plutôt une demande de retrait ou sinon un avis défavorable. Je mais aux voix. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Monsieur de Nicolas il. Le cas dernier. Surveillance fait partie des moyens de lutte contre l'incendie en forêt. Il est donc important de de l'ajouter à la liste des actions à mener dans le cas de la stratégie du développement forestier donc après le mot prévention aussi insérer le mot de surveillance. Madame la rapporteur. Non, mon cher collègue, cet amendement il est satisfaite, puisque nous avons adopté un amendement en commission la semaine dernière, incluant la surveillance dans l'émission incendie des. Stratégie locales de développement forestier donc il est satisfait. C'est donc une demande de retrait. Très bien, je dois l'article 23 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté l'amendement 61 Madame Jourdan. Merci madame la présidente. Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à demander la remise d'un rap. Port du gouvernement au Parlement sur l'opportunité de créer des plans locaux forestier à l'image des plans locaux d'urbanisme à l'échelle des communes ou des intercommunalités. Cette proposition de loi illustre en effet. La nécessité d'adapter l'ensemble de nos documents d'urbanisme au risque incendie. Nous partageons tous cette volonté et nous pouvons également entendre sur le terrain des acteurs locaux réclamer une véritable refonte de notre gouvernance parmi ces voix, certains élus de communes forestières qui préconise de réfléchir à la possibilité de mise en place de plans locaux forestier qui permettrait là mais l'orientation de la gestion et de la prise en compte du risque feu de forêt en repositionnant les élus au coeur des discussions sur l'aménagement forestier globale. Les sénateurs serre estime donc que cette possibilité doit être envisagée sérieusement. Tout en considérant qu'il a pas re-prématuré d'un propose ici d'un, proposer une traduction législative dans le cadre de leur présente PPL PPL sachant que c'est un aveu d'amendement d'appel et que comme tous les rapports sont refusés. Je pense que nous serons appelé au retrait. je salue néanmoins la démarche de ma collègue qui est de, de souligner l'intérêt de cette de ce dispositif que sont les plants forestiers locaux. Qui à mon avis on on. Avenir ou en tout cas mérite que qu'on se penche sur ce sur ces propositions à l'avenir. Ce que nous avons fait quand même en partie sur cette PPL ma chère collègue puisqu'avec le droit de préemption DFCI avec l'inclusion de la DFCI dans les stratégies locales de développement forestier on on avance quand même sur le sujet, mais pour les raisons que vous avez évoqué, ce sera une demande de retrait. Merci. Madame la ministre. Quelques secondes pour compléter. La réponse de Madame la rapporteure donc. Rappeler que le regroupement de la gestion forestière est une priorité du gouvernement dans le cadre de la planification écologique, rappeler que nous avons mis en place un groupe de travail visant identifier les actions à conduire, madame la sénatrice Jourda est que l'instrument plan local forestier va être étudiée dans ce cadre et donc les propositions de ce groupe de travail sont attendues avant l'été. Nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement sinon avis défavorable je vous remercie. M. Jourdas. Je retire donc cet amendement mais à regret parce que je trouve un peu dommageable que chaque demande de rapport soit toujours à à à à assurer d'un avis négatif, c'est vraiment très ennuyeux.

aux ressources forestières et les voies DFCI. Ceci pour maximiser les possibilités d'utiliser des pistes existantes lors des opérations de DFCI, surveillance et luttes dans sa rédaction actuelle l'article IV et trop précis sur le niveau requis organisationnel de participation. L'ONF qui n'est sans doute pas forcément le plus adapté pour une réflexion qui pourra être. L'amendement L'amendement proposé laisse dans sa rédaction plus de possibilités à l'ONF pour le choix de son représentant, tout en insistant sur notre souhait d'avoir quelqu'un de local qui connaissent le territoire concerné par ce cahier des charges.

Oui madame. Ah présidente cet amendement à l'initiative de mon collègue. Franck Menonville éminent agriculteurs vise à inclure les chambres d'agriculture dans l'élaboration du cahier des charges dont le but est d'améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et les pistes de défense des forêts contre les incendies en effet les chambres d'agriculture, de par leur connaissance des voies d'accès au face agricole et boisée dans les territoires sont des acteurs incontournables pour l'élaboration de ce cahier des charges et ses voix étant souvent d'usage partagé entre agriculteurs et acteurs de la forêt. Beaucoup d'agriculteurs utilisent régulièrement ses pistes de défense des forêts contre les incendies et ils peuvent donc apporter une valeur ajoutée certaine en participant clé des charges qui améliorera la mutualisation des voies d'accès. Si le 83. Madame la présidente de la trompe peut-être monsieur Gary là bien défendu. Monsieur Bourgi. En revanche, je ne me paraît. Déterminé à défendre. Madame la présidente, effectivement je vais défendre l'amendement que nous avons cosigné avec notre collègue Jean Jacques Michaud. Madame la ministre Madame messieurs les rapporteurs, vous le savez tous, la chambre d'agriculture est hein d'une chambre consulaire qui tire sa légitimité de la connaissance des territoires et les terroirs qui sont celles de ses ressortissants. J'ai pour habitude de dire que les agriculteurs sont les architectes de nos paysages de nos bocages de nos vignobles et de nos forêts et très souvent lorsqu'il y a des incendies, ce sont les agriculteurs et les viticulteurs qui accompagne et qui guide. les bénévoles des comités comme toi le de faux de forêts qui guide accompagne les sapeurs-pompiers lorsqu'ils interviennent afin de leur montrer de les guider sur ces terrains sur ces territoires et sur ces routes. Que parfois une mais qu'ils ne connaissent pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle nous semble nécessaire et légitime d'avoir la chambre d'agriculture incluse à part entière dans ce dispositif. Alors je voudrais d'abord précisé qu'il s'agit donc des dessertes forestières. Et et qu'il s'agit des dettes lire un un cahier des chartes des dessertes des massifs forestiers de manière à ce que les véhicules. Du SDIS puisse y accéder dans les meilleures conditions et intervenir en cas d'incendie dans le cadre de ce cahier des charges des voies forestières. Nous avons donc proposé d'associer à ce travail de de de rédaction. Les propriétaires forestiers. Et les gestionnaires en fait les financeurs, ceux qui vont financer les travaux qui répondront au cahier des charges. Donc il nous semble pas. Nécessaire d'y intégrer les chambres d'agriculture. Sachant qu'il s'agit donc exclusivement des voies forestières bien sûr tout à l'heure nous avons parler des cartes d'aléas ou des schémas desserte plus globaux. Incluant les espaces naturels ou là bien évidemment, les agriculteurs ont ont toute leur place pour participer au cahier des charges. Voilà, nous pensons qu'il est plutôt. Nécessaire d'éviter une multiplication des acteurs pour ne pas alourdir ses démarches et et ne pas n'auront plus alourdir les coûts de ces dessertes forestières qui sont, je le rappelle quand même déjà très élevés. Et s'agissant des dessertes qui peuvent avoir de multiples riverains par exemple des agriculteurs, je pense que chacun d'entre vous, aujourd'hui il est confronté. Hé bien on a aussi le riverain, en l'occurrence l'agriculteur si il les forestiers, les propriétaires de la forêt de toute façon il sera associé dans le cas de ce cahier des charges. Mais donc on associe l'agriculteur parce que d'abord on on va l'associer à à au financement aussi hein de cette desserte s'il demande à ce qu'il y ait des passages spécifiques pour accéder à ces propriétés. Voilà donc pour toutes ces raisons, mes chers collègues, ce serait plutôt une demande de retrait un avis défavorable puisque je le précise, il s'agit uniquement de cahier des charges des travaux des voies forestières. Dans les massifs forestiers. Un ministre. Claire donc. Demande de retrait sinon avis défavorable pour les mêmes raisons que Madame la rapporteure Gremy monsieur Gremillet pour une explication de vote.

On a vécu et je l'ai vécu dans le département des Vosges, on a six vosgien effectivement on s'est rendu compte avec les incendies. C'est la première fois qu'on avait des incendies de cette dimension. Cette proportion. Que toutes les nouvelles dessertes forestières. N'était pas dans les cartes communales. Elle ne figurait dans aucun document. Forestier. De tout et par rapport au au desserte préexistante au préalable. Et on s'est rendu compte effectivement. Que tout le travail il dépend de la commune. De l'ONF lorsqu'on a dû domaniale mais surtout des propriétaires privés et comme l'a dit notre rapporteur c'est eux qui financent en totalité les travaux de la desserte. Et par contre il est opportun hein. D'avoir une cartographie de ces nouvelles dessertes qui sont d'ailleurs financées par les régions et avec des concours communautaires. Il est intéressant. D'avoir l'avis. Du SDIS par rapport parfois peut-être de prolonger d'une une desserte une piste de quelques centaines de mètres, pour avoir une une accessibilité bien plus grande au Massif qui n'est pas desservi. Et il est aussi. Intéressant de ne pas apporter de surcoût, je partage complètement le propos de 3 porteur ce que ces dessertes sont complètement financée par les propriétaires qui sont concernés et en général il y a pas d'agriculture c'est que du, on est dans le domaine du massif forestier par contre je voudrais en profiter pour dire et rendre hommage au travail qui est fait et les chambres d'agriculture pourrait avoir un rôle mais pas dans ce domaine-là en matière de transport d'eau qui vient à abonder les concours des pompiers. Ça a été fait dans le département des Vosges. Ça a été magnifique et peut-être qu'il y a quelque chose à légiférer là aussi d'. Qui diminuerait les coûts donc je partage l'avis de notre rapporteur sur les dessertes. C'est un autre sujet. Merci je vais donc mettre aux voix ces amendements. Ces quatre amendements identiques qui ont reçu un double avis défavorable qui est pour.

Non. Ce présent amendement. Vise à réduire de 10 à 5 ans la durée de mise à jour du cahier des charges et de la cartographie des. Des Dacr c'est Merci madame la présidente, madame la ministre Madame la rapporteure. L'article 24 prévoit l'élaboration par les SDIS RPF et ONF d'un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et puis de défense des forêts contre les incendies le prévoit également que chaque région devra établir une cartographie de ces voire d'accès et de défense, nous sommes donc favorables bien sûr à cet article. Mais cette cartographie régionale devait être à jour tous les 10 ans. Je tiens à souligner justement au niveau des incendie hors-norme, que nous avons vécu que l'établissement au jour le jour de cette cartographie absolument essentiel, on a vu aujourd'hui des sapeurs-pompiers qui devait être assisté par les locaux par la DFCI local pour pouvoir trouver les chemins d'accès. Or en numérisant. Aujourd'hui on est en capacité de mettre à jour. Pratiquement au jour le jour. Justement c'est vrai d'accès suffit que les DRCI le fasse remonter au niveau régional, donc il n'est pas utile d'attendre 10 ans voire même 5 ans, on a la possibilité d'une mise à jour pratiquement en réel. C'est pourquoi nous proposons que cette mise à jour se fasse de façon constante dès que des évolutions sont observées. Si madame la rapporteure. Quel est votre avis sur le l'amendement. Alors c'est un avis défavorable puisqu'une mise à jour constante nous semble irréaliste d'un point de vue pratique. Madame la Ministre, quel est votre avis sur l'amendement de la commission et celui de Monsieur Alors à la vie sur l'amendement de Madame Loisy est favorable et par contre nous demandons Monsieur Gillet comme Madame la rapporteure de bien vouloir retirer son amendement sinon l'avis est défavorable. Bien je vais donc mettre aux voix, ces deux amendements. D'abord le 138 qui a qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour.

Madame de Marco pour le 126. Voilà c'est une demande de suppression de cet article. Les dispositions prévues par la tique 25 sont déjà satisfaites par l'actuelle rédaction du code forestier, il exclut d'ores et déjà du défrichement les déboisements permettant de créer des équipements indispensables à la protection des forêts il exclut également du défrichement des déboisements destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale et à la mise en valeur d'anciens terrains agricoles ainsi l'article 25 ne constitue pas une avancée en matière de protection des forêts contre l'incendie. Au contraire, l'association de défense de la forêt contre un incendie de Nouvelle Aquitaine, alerte sur le risque de défrichement injustifiée. D'ailleurs le selon le rapport sénatorial sur lequel est basé cette proposition de loi, l'administration et les forestiers sont peu favorables à ce type de mesures. La prévention et la lutte contre les incendies nécessite des aménagements indispensables mais nous ne réduirons pas le risque incendie en coupant la forêt. Merci madame la présidente. Chers collègues Madame de Marco. Vous doutez bien qu'un article de suppression. C'est un amendement de suppression sur un article et maintenant notre proposition de loi n'aura et puis effectivement qu'une demande de retrait ou un avis défavorable. Plus sérieusement. La première mouture de l'article 25 pouvaient à la rigueur souffrir certaines critiques quant à l'opportunité de faire des défrichements abusifs. On l'a resserré en commission de manière justement à éviter cette possibilité. Donc vraiment, on vous demande. Sympathiquement de retirer votre amendement

À l'article 27. Madame la présidente de la. Vous avez un amendement 16. Oui merci madame la présidente. En fait c'est un amendement retex retour d'expérience personnelle que doit-on prendre en cas d'évacuation. Que faut-il absolument avoir sur soi. Si l'on part sans rien. Quels vêtements a minima sur soi. Si l'on a un sac et si l'on peut effectivement évacué à voir avec sa voiture. Ça paraît simple, quand on n'est pas. Confronté. À l'évacuation. Mais c'est un moment compliqué. Et complexe si. Nous ne sommes pas préparés à évacuer. Comme peuvent l'être par exemple, les femmes enceintes à qui l'on préconise un petit bagage et une liste de choses à emporter et je pense qu'il est indispensable que nous ayons cette même démarche que nous puissions savoir quoi emporter que prendre notamment dans les papiers. Des originaux, comme le livret de famille puisque vous savez que ces livrets de famille ne sont pas duplicable ou encore ça peut paraître bizarre, une bonbonne de gaz. Oui, moi j'ai vu pendant ces feux ces incendies des bonbonnes de gaz. Brûlés et agir comme des petites bombes et blessés, nombre de non-, pompiers. Il faut aussi le savoir et s'en rendent contre chaque minute est précieuse dans ces situations d'évacuation d'évacuation. rationaliser ce moment en ayant une liste d'évacuation. Je pense que. Ces gestes ou cette liste des évacuations fait partie des gestes qu'il faut. Apprendre. À nos concitoyens dans. Les moyens de communication qui sont les nôtres et qui vont être les nôtres dans les mois à venir pour préparer la période des incendies de de cet été, merci. Pas de mal, madame la présidente. Chers collègue Nathalie Delattre telle qu'il est rédigé votre amendement insère une fonction de sensibilisation des particuliers aux gestes de sécurité domestique et aux mesures d'évacuation a réalisé en cas d'incendie. Parmi les fonctions des chambres d'agriculture. Il me semble pas que les chambres d'agriculture soient les bons acteurs pour mener ses actions de sensibilisation qui ne sont aucunement porter sur le monde agricole. C'est la raison pour laquelle on émettra un avis défavorable. Madame la Ministre même avis. Je mais aux voix, madame la présidente, qui est pour double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il ne n'est pas adopté l'article 27 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est adopté à l'article 28, un amendement du gouvernement. L'amendement 103 Madame la Ministre. et en indemnisant le cas échéant, les agriculteurs pour les coûts induits hausse de charges récolte détériorer la réglementation des activités agricoles vis-à-vis du risque incendie est déjà possible et pratiqué dans les arrêtés préfectoraux pris en application du elle 131 du code forestier la proposition permet donc de mettre en avant ce type de réglementation et l'ancrer dans la loi néanmoins. S'agissant d'une indemnisation spécifique des agriculteurs. Il peut être considéré que les contraintes sont limitées dans le temps justifié par l'intérêt général et que d'autres professions peuvent également être soumises à ces contraintes de limitation d'activité dans les arrêtés préfectoraux sans qu'il ne soit non plus indemnisés. Par ailleurs, il est actuellement prévu une indemnisation à hauteur des coûts nets induit mais il sera extrêmement difficile de les déterminer. En effet si nous reconnaissons aisément que travailler de nuit plutôt que de jours par exemple est beaucoup plus pénible pour un agriculteur quel en est le coût Net induit. Nous émettons donc un avis. Des la, non c'est c'est c'est notre amendement. Et qui se termine par une question en fait en effet si je reconnais aisément que travailler de nuit plutôt que de jours par exemple est beaucoup plus pénible pour un agriculteur, qu'elle en est le connaître un devis. merci. Alors pour ce qui est de l'avis du gouvernement va solliciter la Commission. La ville l'avis sur l'amendement du gouvernement nous allons solliciter la commission. C'est moi qui vais mettre un avis Madame la Ministre. Merci madame la présidente, madame la Ministre. Si nous avons prévu dans le texte initial une indemnisation des agriculteurs soumis à une obligation de réalisation des travaux agricoles. La nuit c'est surtout dans un objectif d'acceptabilité de cette mesure qui nous semble essentiel à la prévention des incendies, mais qui fait porter de très fortes contraintes, contraintes sur les agriculteurs. C'est pourquoi l'avis sera défavorable à cet amendement de suppression de suppression présentée par le gouvernement. Je rajouterais juste personnellement que, effectivement, faire des travaux, la nuit, ne serait-ce que des récoltes de blé. C'est des fois meilleur la paille et de meilleure qualité et le blé à meilleur PS Si on veut qu'il soit accepté. Il ne faut pas oublier d'introduire la possibilité d'une indemnisation donc avis défavorable. Je mets aux voix c'est un amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'article 28 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est adopté le 133 Madame de Marco. Merci. Cet amendement s'appuie sur la recommandation numéro 46 du rapport sénatorial ayant donné lieu à cette proposition. En effet, à rebours des orientations promis par ce rapport. Un récent arbitrages du gouvernement pénalise fortement le financement par la PAC des peste pratique pastorale d'un temps de lutter contre les incendies en effet pour la nouvelle programmation Pâques les surfaces pastorales sur les territoires les plus difficiles ne recevront plus d'aides directes. Si elle ne respecte pas un changement minimum de l'Hérault le 2 UGB à l'hectare. Je traduis. Unité gros bétail. Cela signifie que les zones de garrigue méditerranéenne et de montagne les élevages plus extensifs avec moins d'animaux à l'hectare ne seront plus considérés comme des activités agricoles et seront brutalement privés d'aide. Il s'agit notamment de ferme qui travaille avec l'eau ONF sur la lutte contre les incendies. De nombreux élus des territoires concernés de tous bords. Politiques alertent depuis des mois le gouvernement sur cette question sans qu'il n'ait infléchi sa position via cette demande de rapport. Nous souhaitons simplement interpeller le ministère sur cette décision incohérente avait la transition agroécologique mais aussi avec le besoin croissant de gestion du risque d'incendie. Merci madame la présidente. Chers collègues de Marco effectivement étant une demande de rapport, ça sera un, une demande de retrait ou un avis défavorable toutefois. Je serais curieux d'entendre la réponse de Madame la Ministre sur ce plancher des vaches. Il serait intéressant de pouvoir avancer sur cette question. Madame la Ministre. Je crois que le rapporteur à solliciter votre vie. Merci madame la présidente. En fait, le gouvernement a porté une attention particulière tout au long de l'élaboration du plan stratégique national sur les dispositions applicables aux surfaces pastorales en particulier. Donc Madame de Marco. En particulier lorsqu'ils ont été régulièrement remis en cause dans le cas des audits européen sur la précédente programmation de la PAC les coefficients d'admissibilité ces surfaces selon la méthode, la méthode dite du prorata qui sous-entendent le niveau d'aide versées sur ces surfaces ont pu être maintenus à un niveau inchangé dans la version finale du PSN adopté par la Commission européenne, ces dispositions permettent de reconnaître l'admissibilité de ces surfaces composée majoritairement de ligne dans plusieurs départements du sud de la France, le maintien de cette méthode du prorata selon des dispositions inchangé a dû s'accompagner de nouveaux critères pour contrôler l'admissibilité de ces surfaces en remplacement des indices de pâturage utilisé sur la programmation antérieures dont la contrôlabilité posaient des difficultés. C'est l'objet du critère de chaud de taux de chargement qui a été introduit pour cette nouvelle programmation et dont le niveau doit être fixé de façon à garantir un entretien par pâturages suffisant ce qui concourt également aux objectifs poursuivis dans le cadre de la lutte contre les incendies en prévenant an fraîchement des surfaces concernées, un taux de chargement trop faible conduirait au contraire à diminuer l'entretien de ces surfaces avec un risque accru en terme d'incendies. Je tiens à souligner par ailleurs que nos nombreuses mesures de la PAC sont favorables au pastoralisme et concourt à maintenir une utilisation effective de ces surfaces notamment le mécanisme de convergence appliqué à l'aide de base. Aux revenus globalement favorable à ces systèmes d'exploitation. L'éco-régime l'aide couplée aux légumineuses fourragères en montagne et le maintien des aides animales maintien d'indemnité compensatoire de handicaps naturels avec un budget préservé, ainsi que le renforcement du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation enfin de mesures agro-environnementales et climatiques visant à l'ouverture des millions tu été spécifiquement créés dans un objectif de défense des forêts contre l'incendie. Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne. Le critère de taux de chargement visés par l'amendement ne s'applique pas pour un certain nombre de dispositifs d'aide listés ci-avant le versement de lycée H, N et des c'est notamment n'est pas conditionnée par ce critère et ce sont ces mesures qui sont davantage conçues pour le maintien de milieu ouvert et donc la lutte contre le risque d'incendie au regard de ces éléments, l'avis du gouvernement est donc défavorable.

Parce que j'ai pas tout noté. Monsieur président retard madame de. Non. Merci madame la présidente. Non mais c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit, je pense, c'est un sujet important sur ce sur ce plafond et on sait qu'on y revient régulièrement, et en tout cas sur la question du du pastoralisme. Et par rapport à ce que vous avez dit effectivement, je pense que là il y a une demande de rapport qui me paraît plutôt bienvenu justement pour pouvoir avancer et c'est c'est exactement ce que vous dites en fait hein pour pouvoir avancer. Sur ces questions là et pour pouvoir trouver une très bonne une trajectoire par rapport à la problématique dont on est en train de de parler donc il, il me semble, pour le coup que. Et je m'appuie sur ce que vous venez dire que la, le rapport est plutôt très justifié. Monsieur Bourgi. Voilà la présidente, je vais intervenir pour appuyer la demande de mes collègues puisqu'effectivement en entendant la réponse de la ministre et j'ai été troublé Madame la Ministre vous le savez bien, en ce moment et depuis quelques semaines, tous les éleveurs dans le sud de la France sur la façade méditerranéenne sont particulièrement mobilisés et inquiet par rapport aux évolutions et aux changements de taux de chargement de la PAC et les réponses que vous avez fait m'interpelle et viennent conforter finalement à la demande de nos collègues du groupe. Écologiste quant à la production d'un rapport, je pense qu'on serait tous et toutes mieux éclairer si un rapport était rendu sur le sujet parce que les propos qui sont portés par les éleveurs et leurs organisations représentatives auprès du ministre de l'Agriculture. Les réponses que vous avez formulé et celle de nos collègues je pense mériteraient qu'on ait un rapport qui permettent d'approfondir la question. Madame la Ministre. Expliquez madame la sénatrice de marque. Échos que. Vous demandez un rapport au gouvernement. On émet un avis défavorable je pense l'avoir motivé vous demander ce rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi sur l'abaissement du taux de chargement minimum. Permettant l'admissibilité des surfaces pastorales aux aides directes de la PAC. Je pense nous avoir clairement répondu dans ma conclusion entre autres sur. Conformément à la réglementation européenne nos critères de taux de chargement visés par l'amendement ne s'applique pas pour un certain nombre de dispositifs d'aide et toutes celles que j'ai listé juste avant. Donc moi je respecte le fait que vous souhaiteriez un rapport nous l'entendons et nous le notons mais nous émettons cependant un avis défavorable. Très bien monsieur le rapporteur. présidente. La présidente, je voulais juste apporter une précision, le taux de chargement minimal dont on parle c'est 0,2. GB hectares. Une brebis, c'est 04. Moi j'ai zéro quatre une brebis avec son agneau une brebis avec son agneau. Je pense que si ce taux. Minimum de chargement été mis par la France. C'est pour répondre uniquement à une demande de l'Union européenne sur les versements de la PAC, mais on est vraiment, c'est le cas de le dire à ras les pâquerettes. Et et je considère, personnellement ça n'engage que moi. Qu'à moins 0, 2 hectares de taux de chargement GB hectares on était plus sûr de l'agriculture mais sur de l'amateurisme et je pense que ça nécessite pas des accompagnement financier de la PAC. Bien. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 133 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui compte. Il s'abstient. Il n'est pas adopté. Après l'article 28, un amendement 132 madame de Marco. Cet amendement s'inscrit dans la lignée du précédent et des recommandations du rapport sénatorial qui a donné naissance c'était de proposition de loi, à savoir la promotion du pastoralisme comme outil de lutte contre le risque incendie 1000 vise cette fois-ci, d'autres outils que les aides directes de la PAC. Il s'agit de proposer via un rapport du au gouverneur du gouvernement au Parlement d'étudier les conditions de développement des mesures agro-environnementales DFCI la mise en place de paiements pour services environnementaux. Lutte contre les incendies, à l'image des paiements pour services environnementaux actuellement développées par les agences de l'eau et qui ont montré leur intérêt. Il s'agit de rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent de la collectivité lorsqu'ils mettent en oeuvre des pratiques durables de gestion du risque incendie sur les territoires particulièrement concernés. Merci. Quelle est la ville de la commission. Madame de Marco. Je partage votre inquiétude sur les mesures agro-environnementales et climatiques. Mais plutôt qu'un nouveau rapport, je vous invite à vous référer aux 975 pages du plan stratégique national de la France qui décline la PAC et retrace précisément les MAEC. Ouverture des milieux. Elle y a l'EMA EC DFCI je pense que vous y trouverez toute la réponse à vos questions et qu'un rapport sera inutile. qui est contre qui s'abstient et n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 29 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté, il est minuit et je vous propose de prolonger notre séance raisonnablement afin d'achever l'examen de ce texte. Tout le monde est d'accord. Alors il en est ainsi décidé à l'article 30. Madame la présidente Delattre. Oui merci madame la présidente, mes chers collègues j'avais posé un amendement qui visait à équiper les. Le professionnel d'extincteurs et qui a été déclarée irrecevable au motif que l'équipement des véhicules relève du code de la route donc réglementaire. Je voulais dire que sur les feux de l'attestent de Landiras hein Nombreux étaient les véhicules professionnels qui était aux abords des lieux de de l'incendie et qui, s'ils avaient été équipés. D'extincteurs aurait pu circonscrire le feu en attendant. Les secours à leur mesure, bien évidemment. Ironie du sort, le. Le véhicule. Qui effectivement est le point d'embrasement et le début l'embrasement du du feu de La Teste était un véhicule professionnel et qui. Était en zone blanche et qui a mis un certain temps avant de pouvoir alerter les secours. Je pense qu'il aurait peut-être pu. Éviter. Un drame s'il avait été équipés d'un extincteur professionnel donc je je déplore les recevabilité je la comprends néanmoins. Je saisirai donc le ministre. Qui est concerné pour une évolution du code de la route. Je vous remercie. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce qui est inscrit dans ses articles 30 et 31 sur la sensibilisation et qui concerne principalement les mégots. L'interdiction de fumer et c'était étaient des choses absolument nécessaire Parfaitement salutaire pour ce projet de loi. Cela dit l'objet de ce titre qui est consacré à la sensibilisation devrait être d'élargir au maximum nos campagnes de prévention afin qu'elle soit présente tout au long de l'année dans la vie quotidienne des Français. Et comme nous savons que 95% des départs de feux sont d'origine humaine et sont souvent accidentelle. Il faut donc s'attacher à développer tous les types de préventions possibles pour que la population puisse acquérir rapidement les bons réflexes. Pour ce qui concerne la sensibilisation. Ce qui serait tout à fait pertinent, ce serait des d'inscrire dans le code de l'éducation comme un amendement de ma collègue Gisèle Jourda le proposera tout à l'heure. Ceci dans le code de l'éducation afin de de former. Tous nos jeunes au risque de prévention d'incendies. En effet, comme tout ce qui touche à la protection de l'environnement, il est indispensable d'alerter le plus tôt possible les jeunes générations sur l'importance des risques auxquels sont exposés aujourd'hui de nombreux massifs forestiers et plus généralement de nombreuses régions touchées par la sécheresse particulièrement sévère cet été et même cet hiver. Une autre de mes propositions consisté à rendre obligatoire des affichages de consignes de sécurité prévention prévention du risque incendie dans les logements de tourisme situées dans les zones particulièrement exposées. Cette proposition a été rejetée par la commission jugée irrecevable article 41 réglementaire. Ce que je conçois, dont acte, tout de même nécessaire que l'on se préoccupe de tous ces petits problèmes matériels comme nous l'avons déjà. Évoqué plusieurs fois car une bannière, d'une manière ou d'une autre, il nous faut aller beaucoup plus loin. Car si les populations du sud de la France ont conscience depuis longtemps du risque incendie. C'est loin d'être le cas ailleurs on parle dorénavant du risque incendie pour la Corrèze où la Sologne, ce qui était inconcevable. Auparavant, les populations de ces territoires ne sont donc pas aussi conscient des conséquences dévastatrices pour la végétation période de sécheresse. Merci. Nous allons maintenant passer l'amendement 136 de Madame de Marco. Avant tout, je tiens à rappeler que des actions de communication pour prévenir l'abandon des mégots dans les territoires exposés au risque d'incendie est une initiative que nous soutenons fortement au sein du groupe écologiste. Leur intérêt majeur d'un point de vue environnemental, économique et social. Elles ont une utilité publique indéniable. Ce que nous souhaitons amendé n'est donc pas l'objectif même de l'article mais plus le moyen pour y parvenir, c'est-à-dire son financement. reste du rédaction actuelle. L'article 30 prévoit de s'appuyer sur la filière de responsabilité élargie du producteur pour financer des actions de communication. Mais cela ouvrirait une brèche dans le fléchage des contributions des acteurs des filières REP ce qui n'est pas souhaitable. Les filières REP ne peut peuvent paître une variable d'ajustement. Nous proposons donc ici une solution alternative plus adapté à ce type d'initiative et qui évite d'impacter les collectivités qui ont besoin des contributions financières des steaks organisme. Pour assurer leur service public de gestion des déchets sans grignoter leur budget. Il paraît logique que des actions de communication sur les listes risque liés aux mégots soit financée par les producteurs de tabac eux-mêmes ceux à qui incombe la responsabilité et par ailleurs, les sociétés privées et très lucrative. Merci. Quel est l'avis de la commission. Merci madame la présidente. Je constate que cet amendement déposé par Madame de Marco. Ne remet pas en cause le coeur de la proposition à savoir faire financer des actions de communication sur le risque incendie par les producteurs de tabac. Sur le fondement de la Cet amendement propose toutefois d'inscrire cette obligation d'or de l'arrête et donc en dehors du cadre législatif à faire en cette solution me semble peu satisfaisante juridiquement par ailleurs consacrer une part des contributions financières des campagnes de prévention ne serait pas un manque à gagner pour les collectivités territoriales comme l'avance l'objet de l'amendement en effet une partie des fonds de la Rep mégots vice-déjà à faire de la sensibilisation sur l'abandon des mégots. Il s'agit par cet article de préciser que cette sensibilisation doit tout particulièrement être mises en oeuvre dans les territoires réputé particulièrement exposés aux risques d'incendie, et dans les bois et forêts classées à risque d'incendie. Vous l'aurez compris, c'est une demande de retrait ou à défaut chers collègues un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice de. En fait nous partageons totalement l'objectif de cette proposition, mais celle-ci est d'ores et déjà en Oeuvres puisque l'arrêté ministériel qui précise le cahier des charges de cette filière prévoit explicitement de de telles actions de communication et de sensibilisation. Les actions de communication doivent notamment informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon nos mégots dans l'environnement ainsi que les sensibiliser sur le risque d'incendie lié à l'abandon de mégots dans l'environnement. En application de cet arrêté publié en décembre dernier, l'éco-, organisme doit également soutenir les collègues. Activités territoriale et le regroupement pour leurs actions d'information et de sensibilisation. nous apparaît que l'objectif de votre amendement est satisfait. Nous invitons à le retirer à défaut de quoi, nous y serons défavorables. Je vous remercie. pour et contre qui s'abstient-il être adopté après l'article 31. Un amendement et un sous-amendement l'amendement 107 et présenté par le gouvernement. Il est défendu.

qui se sont déroulés en métropole l'été dernier, ainsi que leur impact sur les acteurs de la lutte incendie comme sur les habitants ont rappelé l'importance de former, d'informer les populations au risque cet enjeu se pose avec une acuité d'autant plus importante que l'évolution du climat accentuera la fréquence et l'intensité de ces feux hors norme mais aussi de toute autre phénomène entraînant la survenue de crises. C'est dans ce contexte que le plan d'action tous résiliant face au risques élaboré à partir des conclusions de la mission culture du risque diligentée par le gouvernement a dessiné plusieurs axes de travail visant à renforcer la sensibilisation des populations face aux risques majeurs et à leur manifestation catastrophe naturelle accident industriel. L'un des objectifs est d'organiser sur l'ensemble du territoire national métropolitain et outre-mer des actions de sensibilisation et de préparation de la population à ces événements pour lesquels le code de l'environnement instaure le droit à l'information des des citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés est également essentiel de former la population française aux bons comportements à adopter en cas de survenue d'un événement majeur pendant et après la crise cette compétence relevant du ministère de l'Intérieur, il est en effet indispensable de connaître la signification d'un signal d'alerte les gestes réflexes à acquérir pour se mettre à l'abri de l'aléa ou de la menace selon la nature de ces derniers et de savoir se préparer dans de bonnes conditions à une décision éventuelle d'évacuation de confinement, le développement d'un citoyen acteur de sa mise en sécurité et de la protection d'autrui se comprend dans la complémentarité du volet formation à la prévention des risques et au comportement en cas d'événement et du volet d'une journée nationale de sensibilisation et de prise de conscience collective des enjeux l'article prévoit donc la création d'une journée annuelle de la résilience face aux risques organisé chaque année le le 13 octobre au moment de la journée internationale de la prévention des risques de l'ONU ainsi que la mise en place d'actions dédié d'information dans les administrations publiques, les établissements et entreprises privées ou les entreprises. l'établissement d'enseignement. Il prévoit également des dispositions. Pour modifier le code du travail pour permettre la sensibilisation de tous les salariés au sein des entreprises. Je vous remercie. Madame, monsieur, rapporteur. Vous avez un sous-amendement présenté à l'amendement du gouvernement en même temps vous donnerez votre avis. Merci madame la présidente. Consiste à supprimer les alinéas 6 avant de ce que vient de proposer, Madame Madame la Ministre. Si je soutiens la pérennisation et l'inscription dans la loi de l'organisation d'une journée nationale de la résilience, qui a lieu, vous l'avez rappelé chaque année le 13 octobre depuis maintenant 5 ans, il ne me paraît en revanche pas c'est tout souhaitable de faire peser sur les employeurs des obligations nouvelles qui s'ajouteraient aux normes déjà en vigueur en matière de sécurité au travail. Je souligne à ce titre que le nouvel article L. 731 1 2 du code de la sécurité intérieure telle que proposée par l'amendement du gouvernement imposerait une obligation d'information sur tous les employeurs sans aucun seuil. En outre, aucune raison ne justifie que la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques. Autre que ceux liés à l'environnement professionnel repose sur ces mêmes employeurs. C'est pourquoi je donnerai un avis favorable à l'amendement du gouvernement sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement qui supprime les obligations reposant sur les employeurs. Madame la Ministre quel est votre avis sur le sous-amendement que vient de présenter le rapporteur. Merci madame la présidente. Donc sur le sous-amendement au 107 que je viens de vous proposer. On peut noter que le conseil d'orientation des conditions de travail et la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle, ont été consultés par la direction générale du travail pour vous rassurer monsieur le rapporteur. Ça veut dire que vous émettez un avis défavorable au sous-amendement du rapporteur. Je suis désolée moi je voudrais je vous demande un avis favorable défavorable ou ça vous avez raison, nous demander Anne. Oui, j'ai aussi la possibilité d'hésiter et de réfléchir. Excusez-moi vous de l'heure tardive mais je maintiens effectivement notre amendement telle qu'il était au départ. Donc c'est un avis défavorable sur le sous-amendement du rapporteur oui madame la présidente. Voilà c'est ce que j'ai besoin de vous entendre dire, madame la Ministre

Madame la ministre je je suis actuellement rapporteur sur un rapport de la délégation aux affaires aux entreprises qui traite justement de la simplification des normes et des règles pour les entreprises. Et ce qui ressort sans livrer ce qu'on va présenter mi-juin sur ce rapport. Mais une des choses qui ressort de façon très importante, c'est qu'on ne devrait plus jamais légiféré sur une nouvelle règle aux nouvelles normes qui s'appliquent à nos entreprises, sans une étude d'impact, voire même un test PME. C'est la raison pour laquelle. Je ne peux moi soutenir un amendement qui entraîne une nouvelle règle aux nouvelles normes aux entreprises sans avoir fait ne serait-ce qu'une étude d'impact qui chiffrent. À la fois en termes de temps, mais aussi en termes d'argent, ce qui serait impliquée davantage aux entreprises. Donc je soutiendrai je voterai dès demain le sous-amendement de mon collègue, Martin. Oui merci madame la présidente, madame le Ministre. Mesdames et messieurs les rapporteurs en soulignant tout le travail que qui a été fait par. Par la la mission. Mais en revenant enfin tous les amendements sont importants. Concernant. C'est important de sensibiliser, faire connaître et cetera. Les dangers les menaces. En particulier dans tous les départements qui ont été concernés tous les collègues. L'ont rappelé. Même si les Ardennes, on était beaucoup moins concernés. On salue où va. Vraiment tout ce qui a été fait et c'est vrai que. Je dirais. Alors concernant cette journée nationale de de de c'est vrai que moi moi dont les Ardennes. Je n'ai pas trop entendu parler. Et bon à coup sûr, c'est important de, de sensibiliser tous les publics. Alors de l'autre côté. Je crois que. Ça a été aussi largement évoqué. Quant à la sécurité. Des personnes et des biens. Bon il y a les communes en général sont dotés de plans communaux de de sauvegarde en liaison avec l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales de tous les partenaires, donc ça c'est aussi un point sur lequel c'est important localement du travailler sans oublier aussi toutes les entreprises comme ça a été rappelé mais. Je soutiendrai le sous-amendement du rapporteur je crois qu'il l'a argumentée

Très bien je n'ai plus de, tu. Explications de vote. Je vais donc d'abord mettre aux voix le sous-amendement du rapporteur qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour le sous-amendement. qui est contre. Qui s'abstient il est adopté, je mets maintenant aux voix l'amendement du gouvernement. Qui est ainsi sous-amendé qui est pour. qui s'abstient. L'amendement est adopté. Ainsi sous-amendé Oui merci madame la présidente, je, je prends la parole sur article puisque j'ai déposé un un amendement qui a été réputé irrecevable. Parce que concernant le code de la route donc réglementaire. C'est un combat que je mène depuis longtemps. Depuis que vous avez vu disparaître les cendriers dans les voitures neuves. J'avais en 2019 alerter le gouvernement dans une question écrite sur les nombreux départs de feu qui sont causés par les mégots que l'on jette par les les fenêtre s'des voitures. Et on m'avait répondu à cette époque. Cela aller si l'on. N'aller dans mon sens, de remettre d'obligée de remettre des cendriers dans dans les voitures, que le message envoyé à la population serait contre-productif, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. Donc je pense que bon ce n'est en rien lié. Avec la prévention. De lutte contre le tabac. Mais je pense que obliger les constructeurs. À remettre des cendriers alors qu'aujourd'hui ils sont soit payants en option soit au pire il n'y a rien. On sait aussi que. Les chewing-gums hein qui sont très longs à être détérioré sont jetés par les fenêtre parce qu'il n'y a plus de 2 cendrier notamment donc je pense que c'est une mesure de bon sens, je regrette qu'on n'ait pas pu la garder encore une fois je je comprends l'recevabilité puisque c'est réglementaire, donc je me fendrais encore d'un courrier auprès du ministre concerné pour faire tenter de faire évoluer la réglementation et de lutter contre le lobbying puissant. Des constructeurs automobiles. Merci madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le rapporteur. Je nous tenions à déposer un amendement qui nous semblait important concernant la reconnaissance du statut des psychologues des SDIS pour faciliter encourager véritablement le recrutement donc là également cet amendement n'a, n'a pas pu être déposées pour des raisons. Réglementaires. Donc je voudrais Madame la Ministre, attirer votre attention parce que la situation est complexe et peu claires, des unités de secours psychologique ont progressivement été mis en place à l'initiative des SDIS depuis le début des années 90 mais leur développement et donc freiner parce qu'il y a pas de clarté et de reconnaissance des statuts des professionnels de la santé mentale au s'investisse un rapport le le faisait remarquer de la commission des lois, le statut juridique des psychologues au sein des SDIS c'est flou mais une majorité d'entre eux sont recrutés en tant que sapeur-pompier volontaire expert mais cet engagement est proche de l'altruisme et et ça pose quand même question par rapport à une forme de professionnalisation au sein des SDIS d'autres psychologues sont côtés en tant que fonctionnaires territoriaux, mais sur la base d'un concours qui ne tient pas compte des spécificités de leur profession. nous sommes tous conscients que les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont soumis à haut niveau de stress des situations très importante psychologiquement. Nous l'avons vécu effectivement en Gironde. Il faut donc absolument permettent leur accompagnement et les USP sont justement là pour ça donc j'attire votre attention sur le fait qu'il serait souhaitable qu'ils soient intégrés dans le corps d'emplois dans la catégorie d'emploi de catégorie A au sein des SDIS pour cette reconnaissance. Merci. Merci. Nous avons un amendement 15 monsieur bureau quoi. Oui merci madame la présidente. La canicule et la sécheresse, soit mis en avant pour expliquer les feux de forêt. Mais un autre facteur joue un rôle crucial, activités humaines. 90% des feux de forêts sont d'origine humaine volontaire ou dans. Cet amendement viennent donc compléter l'interdiction de fumer. En prévoit il y a également de ne pas allumer de feux aux abords des forêts ou de la végétation, quel qu'en soit la forme barbecue par exemple très pratiqué dans nos régions Mireille méridionale où la raison. Telle est l'objet de cet amendement.

à toute personne autre que le propriétaire d'un terrain de porter ou d'allumer du feu sur ce terrain si est situé dans un bois ou une forêt ou s'il est situé dans le périmètre de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt. Vous avez demandé donc. Le retrait ou un, ou un avis défavorable. Comme ce soir dans cette et Mexique. On est très sage, je vais suivre leur apporter on administre je retire mon amendement. Bien nous avons un amendement 139 du rapporteur qui est un amendement de coordination logistique si madame la ministre, n'y voit pas d'inconvénient. Aucun. Donc personne ne s'y oppose non plus. Il est donc adopté alors là je me vois l'article 31 qui est pour. Et contre qui s'abstient il est adopté après l'article 31. Madame la présidente Delattre. Pour un premier amendement.

contre les incendies dans ce cadre, ils sont amenés à sensibiliser la population, et également à superviser des travaux d'aménagement de prévention. Cela étant, je pense qu'au-delà de la seule prévention et sensibilisation leur présence sur le terrain pour être rendu plus efficace en inscrivant ses agents comme personnel habilité habilité à constater les infractions forestière notamment pour protéger les pistes et infrastructures structure pardon DFCI des infractions qu'elles peuvent connaître. Je vous remercie. Merci madame la présidente. sur les voies, DFCI les dépôts sauvages d'ordures augmentent l'Exposition au risque de départs de feux d'espaces forestiers il donc nécessaire d'améliorer le dispositif de surveillance en élargissant le périmètre de compétence des agents assermentés qui interviennent dans la surveillance espaces forestiers. Cet élargissement concerne uniquement les agents opérationnels. Les agents de droit public droit privé des structures de défense des fois quand tu l'incendie sont déjà chargé de la prévention des feux de forêt. Ils sont amenés dans le cadre de leur travail à sensibilise la population et supervisé les travaux d'aménagement. Il contribue à prévention des incendies dans les massifs forestiers qui peuvent avoir un effet dévastateur sur les espaces naturels ainsi pour protéger les pistes, les infrastructures de la DFCI, cet amendement vise à habiliter les agents de droit public et de droit privé des structures de défense des fois quand l'incendie à constater les infractions forestière. Merci madame la présidente. Donc sur ces deux amendements identiques. Quick, 28 et 35 rectifié. Il me semble disproportionné de confier aux agents des Zaza 2 DFCI qui je le rappelle sont des associations de propriétaires, une mission de police. Je demande néanmoins l'avis du gouvernement sur ces deux amendements pour qu'il puisse nous éclairer sur leurs implications juridiques et sur le nombre de personnes qui pourraient être concernées. Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Mesdames les sénatrices la Sarah des de Lattre. Et monsieur le rapporteur. Donc votre amendement mesdames propose d'inscrire les agents des associations syndicales autorisées. Les Zaza chargé de la prévention des feux de forêt comme personnel habilité à constater. Les infractions forestière si nous comprenons la je vais l'objectif de cette proposition, augmenter la force de dissuasion dans les feux dans les forêts à risque, il interroge sur le fond et sur la forme, sur le fond les hasards sont pour l'essentiel, composée d'agents bénévole assermentés uniquement les agents contractuels n'aurait que peu d'effets sur le terrain. Or il n'est pas possible d'envisager d'assermenter des agents. Bénévoles sur la forme, le texte est beaucoup trop vaste car il vise tous les personnels des Zaza partout en France. Par ailleurs, il ne parle pas du commissionnement en préalable à l'assermentation comme c'est le cas dans l'article L 161 tiré quatre que vous indiquez. Lequel stipule commissionné à raison de leur compétence en matière forestière et assermentés à cet effet. En l'état. L'amendement pose beaucoup de difficultés pour ces raisons je vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, nous émettrons un avis défavorable. Merci. Donc métro voit ses amours et vous leur direz aussi madame la Sarah. Vu les explications de Madame la ministre et du rapporteur. Je suis d'accord pour le retirer. Madame Jourda l'amendement 72. madame milite Madame la Ministre, mes chers collègues, nous abordons ici un autre aspect de la lutte contre les incendies, à savoir la sensibilisation des plus jeunes sur les risques actuels, les comportements à adopter ce à éviter. Nous savons tous que les bons réflexes s'acquiert au plus jeunes et qu'à l'inverse, il est parfois difficile de s'en affranchir avec le temps. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de compléter l'enseignement dispensé lors de la Journée défense et citoyenneté par une sensibilisation aux risques incendie. Nous visons cette journée car tous les Français recensés sont tenus d'y participer, ce qui permettrait une couverture très large, il ne revient pas à la loi d'un définir le contenu, les elle pourrait porter à la fois sur les feux de forêt mais également sur tous les autres feux de VG de végétation mais également sensibiliser sur les comportements du quotidien à risques particulièrement d'un certain territoire à haut risque d'incendie ou le moindre mégot de cigarette par exemple peut déclencher une série de catastrophes Je vais avec l'autre parce qu'il est tout à fait complémentaires mais il cible une autre donc. Un autre public jeune pour sensibiliser au risque incendie. de compléter l'enseignement moral et civique dispensé au collège et lycée par une sensibilisation aux risques incendie. Nous avons bien conscience que le Champ des enseignants. Des enseignements dispensés ne cesse de croître ces dernières années au travers des différentes lois que nous examinons au Parlement. Toutefois, dans certains territoires, le risque incendie est omniprésent et il nous sommes dans nécessaire d'informer et de former au mieux nos enfants qui seront les futurs citoyens engagés responsable de demain que ce soit dans les collèges et lycées où il y a des journées prévue pour l'évacuation en cas de risque cet enseignement complémentaire serait le bienvenu. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements. 72 73. Merci madame la présidente. Tout d'abord sur l'amendement 72 concernant la la. Prévention du risque incendie lors de la Journée défense et citoyenneté. Votre votre amendement est justifiée par l'objectif que je partage de sensibilisation des jeunes adultes au risque incendie. Nous devons néanmoins faire preuve de réalisme quant au caractère limité de la Journée défense et citoyenneté, laquelle ne dure comme son nom l'indique qu'une seule journée. Or la liste des thématiques qui évoque l'article L 114 3 du code du service national que vous souhaitez compléter et des jalons, je cite, égalité entre les femmes et les hommes. Lutte contre les préjugés sexistes information sur la prévention des conduites à risques pour la santé. Information sur le don d'organes. Présentation des objectifs généraux de la défense nationale et caetera et caetera. Soyons lucides, si votre amendement est adopté, il ne se matérialisera que dans la. La consécration La consécration de quelques petites minutes sur les thèmes des incendies dans une journée au cours de laquelle les participants sont déjà fortement sollicités, au risque de les saturée d'informations en outre votre amendement est partiellement Satish puisque ce même article L. 114 3 imposent déjà une présentation je cite là encore du modèle français de sécurité civile et des possibilités d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, je note que le dispositif de votre amendement est beaucoup plus large que son objet puisqu'il concerne tout type de feu et non les seuls feux de forêt et de végétation pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable sur cet amendement concernant l'amendement 73. Qui lui. Intéresse la formation des élèves cet amendement qui vise à intégrer explicitement la prévention au risque incendie dans la formation des élèves va à l'encontre de la position exprimée par le Sénat, lors de la récente adoption du rapport de la mission d'information sur la redynamisation de la culture citoyenne. Ce rapport, adopté à l'unanimité des membres de la mission d'information dont votre groupe a notamment rappelé qu'il ne relevait pas du rôle du législateur d'écrire les programmes et a recommandé d'assurer la stabilité du socle juridique de l'enseignement moral et civique. Je note par ailleurs que votre amendement est partiellement satisfait par l'article L. 312 19 qui prévoit déjà une sensibilisation des élèves à l'environnement à la connaissance et des savoirs relatifs à la nature à la nécessité de préserver la biodiversité à la compréhension et à la validation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. Je vous propose par conséquent de faire confiance à la liberté pédagogique des enseignants en retirant cet amendement avis défavorable également sur cet amendement 73. Ministre. Même même avis sur les maisons, 12 et 73. Bien je vais donc les mettre aux voix d'abord le 72 ou Baby défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 73 même vote. Même vote après l'article 31. Nous avons.

des campagnes annuelles obligatoires dans les médias sur le risque incendie puisque nous savons 90% des feux sont d'origine humaine. Ces campagnes nationales de sensibilisation doivent mobiliser des supports variés, allant des programmes scolaires aux campagnes d'affichage en passant en moyenne en parler des par les réseaux sociaux et pourquoi pas une sorte de météo des forêts à l'image de la météo des plages. Elles doivent être renforcées, ne pas se limiter à la période estivale, la prévention, nous considérons et l'affaire de tous. C'est le sens de notre amendement. Oui il est pratiquement identique. Il a été très bien défendu. Je vous remercie. L'avis de la commission sur ces deux amendements. Merci madame la présidente. L'avis sera défavorable sur ces deux amendements. Non seulement parce qu'ils sont satisfaits, puisqu'une campagne de sensibilisation a lieu déjà chaque année depuis 2018 mais aussi parce que je pense que la liste des participants à cette campagne de sensibilisation doit rester souple pour s'adapter aux besoins constatés chaque année.

qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le. 100. Même vote même. Après l'article 31. Madame de Marco le 125. 125. Je vous remercie. La restriction d'accès aux massifs forestiers sont des mesures de prévention efficace. Lorsque le risque incendie est élevé, mais en dehors du Sud-Est. Ces mesures sont peu ou mal utilisé. Donc c'est une demande donc de rapport qui vise à étudier l'opportunité de restreindre l'accès aux massifs forestiers dès que le risque d'incendie est élevé ailleurs que dans le Sud-Est par exemple. Monsieur le rapporteur. Merci à vous. L'article L 131 6 du code forestier permet déjà aux préfets dans chaque département de restreindre les accès aux massifs en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé la demande de rapport me semble donc satisfaite c'est demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Il est retiré. Le 78. Madame Préville. Merci madame la présidente, madame la Ministre Michard collègues. Cet amendement vise à rendre éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local a décile et services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS en effet sa dotation n'est pour l'instant vous le savez réservé qu'aux communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. les SDIS peuvent être propriétaire de caserne. C'est le cas par exemple du SDIS du Lot, propriétaire de la caserne de Cahors. Elle est malheureusement obsolète très mal situé, il y avait donc nécessité de reconstruire une nouvelle caserne à un autre endroit. Oui mais. Puisque c'est le SDIS de Cahors qui est propriétaire, pas de possibilité d'obtenir une subvention de l'État. Pour un service public indispensable à la population est particulièrement aujourd'hui où le risque d'incendie augmente. C'est difficile à concevoir et d'une certaine manière très peu logique j'alors interrogé le prof. Le préfet en lui demandant s'il y avait possibilité de dérogation. La réponse fut négative ai à leur poser une question orale et le ministre Joël Giraud ça s'avéra très très positif en m'indiquant comment on devait procéder pour mener à l'obtention de cette des qui a été finalement obtenu pour 2 millions d'euros. Donc voilà pour éviter peut être que d'autres cas se présente. Je pense que ce serait bon d'inscrire quand tu les SDIS sont propriétaire des casernes qu'qui puisse avoir droit à des subventions d'État, ça me paraîtrait tout à fait logique. Voilà. Cursus L'amendement de de Madame Préville pose un constat. Qui est celui de la nécessité de trouver de nouveaux leviers d'investissements pour les 10 établissements publics. Mais je demanderai le retrait de votre amendement pour plusieurs raisons, chers collègues. Il me semble tout d'abord que les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déjà bénéficier dans certains cas de subventions Titre de la décile et plus particulièrement lorsque cette subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le préfet. D'autre part votre amendement pourrait être en août conduire un saupoudrage des investissements et impliqué des effets d'éviction sur les financements des projets des collectivités locales. Dans la mesure où l'ouverture de la déciles au SDIS n'impliquera pas nécessairement une augmentation de cette enveloppe. Je rappelle également qu'une dotation spécifique de soutien à l'investissement des SDIS existent déjà et fait l'objet d'un renforcement dans le cas de la dernière loi de finance, puisqu'elle a été porté à 150 millions d'euros sur 5 ans. En tout état de cause, il me semble que ce sujet aura davantage sa place dans les discussions sur notre prochain projet de loi de finances 2024. Vous l'aurez compris, c'est une demande de retrait et à défaut un avis défavorable. Le ministre.

que si elle veut effectuer des travaux sur ceux-ci alors. Elle bénéficie de ces dotations si la maîtrise d'ouvrage est assurée par le This. Le projet n'est en principe pas éligibles comme cela vient de vous être 10 cependant des dérogations sont néanmoins prévues par le CG Et en 2021, ces 3 SDIS qui ont directement perçu de la déciles pour un peu plus de 700.000 euros. Mais il ne nous semble pas utile pour les raisons indiquées par monsieur le rapporteur de prévoir d'aller au-delà de ses possibilités. Rendre éligibles de droit, les SDIS à la décide conduirait à la détourné de son objet qui est de financer les projets d'investissement porté par le bloc communal. Je voudrais rappeler, comme cela vient d'être dit que en 2023 donc le pacte capacitaire est porté à 180 millions d'euros 150 plus 30. plus 30. Pacte capacitaire destiné à financer de l'investissement. Pour les SDIS. Bien je vais mettre aux voix Steinman dans 78 qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le sang hein madame variable. Oui. Il s'agit là de prendre en considération la valeur du sauver pour mieux calibrer les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. C'est ce qui ressort en tout cas des de mission parlementaire sur la prévention des risques, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ce calcul de la valeur du sauver permettrait une valorisation de l'action des secours en calculant la valeur des biens qu'ils ont réussi à sauver lors d'un sinistre grâce à leur intervention. Cela permettra aussi de montrer que les dépenses publiques qui leur sont accordés représente un choix d'investissement efficient cette évaluation permettrait une comparaison avec les montants déployés en matière de lutte et de prévention et inciterait au développement d'une politique de défense contre les incendies plus ambitieuse. Particulièrement dans les territoires où la forêt n'est pas ou peu valorisé économiquement de plus lors de la présentation du rapport de la mission de contrôle. Il a été rappelé que le succès de la stratégie nationale et interministérielle, proposée par la présente, proposition de loi reposera sur une amélioration des connaissances et des données relatives aux feux de forêt et de végétation ainsi que sur la nécessité de mieux évaluer la valeur du sauver soit la valeur de ce qui peut être sauvé en cas de sinistre, autrement dit les coûts évités par les politiques de lutte et de prévention. C'est pourquoi il nous sommes nécessaire d'avoir une méthodologie claire d'évaluation de la valeur du sauver et c'est le sens de notre amendement. Chers collègues. Je vais demander le retrait de cet amendement. Bien que je partage votre constat sur cette question qui est et qui revient régulièrement désormais depuis quelques années sur la nécessité d'une meilleure prise en compte de la valeur du sauver dans le calibrage des moyens de prévention et de lutte contre les incendies. Toutefois, il ne me semble pas opportun de multiplier les demandes de rapport au gouvernement. En outre, la rédaction de votre amendement ne me semble pas totalement satisfaisante puisqu'elle laisse supposer que le rapport. Doit uniquement se concentrer sur les moyens de lutte et plus particulièrement sur les financements des SDIS alors que notre rapport d'information du mois de d'août dernier proposer également des temps cette méthodologie pour calibrer les moyens de prévention s'éteint global, c'est la prévention et on pourrait même y mettent la prévision le le volet opérationnel ce sera donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable mais je souhaiterais tout de même que le gouvernement nous expose son point de vue sur cette question qui me paraît importante demande de retrait à des fois un avis défavorable Merci madame la présidente, madame la sénatrice var Elias. Monsieur le rapporteur. Nous partageons votre intérêt sur la mise en place d'une méthodologie claire sur la valeur du sauver. Nous différons toutefois sur l'intérêt du rapport que vous proposez. En effet, le ministère de l'Intérieur des Outre-mer travaille à la mise en place d'une telle méthodologie national ces travaux à forte dimension interministérielle nécessite toutefois une large concertation sur une durée importante afin de disposer d'une masse critique de donner au vu de leur généralisation. Le délai de six mois ne permettra pas de répondre aux objectifs attendus et de produire un travail de qualité que nous jugeons nécessaires, donc nous vous demandons, comme monsieur le rapporteur. Le retrait de votre amendement. À défaut, nous nous émettrons un avis défavorable. Tiens je. Mais cet amendement 5 doubles Avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois l'article 32 qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Article 33 même vote. Même votre article 34 même vote. Même vote adopté. Nous passons après l'article 34 à un amendement 20 de madame Delattre. mais aucun mort. Nous le devons à l'excellence du travail des pompiers et vous nous vous le devons aussi à une politique de prévention. Du à de nombreuses évacuations. Ordonnées par Madame, la préfète de région et sur des périmètres conséquent. Qui ont eu des impacts sur la vie économique locale et à l'heure de se tourner vers les assurances il y a eu des soucis même de gros soucis puisque beaucoup d'assureurs n'ont pas pris en charge les pertes d'exploitation. Pourquoi parce que. Ils n'ont pas été touchés directement par le sinistre. Beaucoup de ces entreprises. Ont été effectivement à plus de 300 mètres du feu et heureusement ils n'ont pas effectivement a été détruit par le feu, mais on leur reproche de ne pas avoir été détruits par le feu, les assurances explique que cela ne rentre pas dans leur clause. De contrat donc c'est plutôt un amendement d'appel. Pour signaler cette aberration parce que. Il faudrait. Comprendre dans les contrats d'assurance que quand ces périmètres sont fermées par décision administrative, hé bien il y a possibilité par pour les assurances de prendre il y a même obligation de prendre en charge les pertes d'exploitation. C'est pourquoi j'ai souhaité ce soir vous présenter cet amendement merci qu'est la ville la commission. Merci madame la présidente. Il sera proposé un avis défavorable à cet amendement qui ne me semble pas satisfaisante tant d'un point de vue. De l'opportunité même que d'un point de vue de sa rédaction. Tout d'abord le dispositif proposé par cet amendement. Semble quelque peu imprécis, notamment en ce qui concerne la notion de décision administrative prise en prévention des risques d'incendie qui ne permet pas d'identifier clairement les cas de figure visé par le dispositif par ailleurs. Il me semble excessif. D'introduire une obligation des assureurs à indemniser les propriétaires pour une perte d'exploitation qui résulteraient non pas de la matérialisation directe et concrète d'un risque mais d'une décision préventive de l'administration. Donc il vous est proposé un retrait ou à des fois un avis défavorable. honnêtement. Sur la disproportion quand vous avez une fleuriste qui ne peut pas venir arroser ses fleurs parce que nous avons été évacués, 10 jours et qu'on lui répond qu'effectivement il aurait mieux fallu qu'elle brûle pour avoir une indemnisation charte sur la perte d'exploitation, alors que effectivement elle n'a pas eu la possibilité d'aller arroser ses fleurs. C'est vrai que je ne pense pas que ça soit disproportionnée c'est juste pragmatique.

Qui est contre

Cet été, on a fait la malheureuse expérience de constater que un certain nombre de sapeurs-pompiers volontaires ne pouvait pas se rendre indisponible par du, du fait de leur employeur. Et donc, l'objectif de cet amendement c'est de, de créer un congé spécial supplémentaire comme il en existe dans d'autres corps pour les sapeurs-pompiers volontaires qui servent dans les territoires réputé exposés au risque incendie incendies, pour éviter qu'il ne, qu'il ne, qu'il puisse ne pas être disponible. Merci monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Il sera demandé à le retrait de cet amendement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne me semble pas. Opportun de créer un congé spécial uniquement réservé aux sapeurs-pompiers volontaires située dans les territoires exposés au risque incendie votre amendement introduit une différence de traitement injustifiée que les sapeurs-pompiers volontaires des autres territoires qui peuvent être légitimement mobilisés pour des interventions en cas de matérialisation de risques d'un autre type. D'autre part s'éteindre cet amendement ne s'inscrit pas dans l'esprit de l'article 34 de notre proposition de loi qui vise plutôt à inciter les employeurs à recruter des sapeurs-pompiers volontaires et à les libérer volontairement il pourrait même avoir l'effet inverse à l'objectif recherché en dissuadant les employeurs de recruter des sapeurs-pompiers volontaires en amont pour ces raisons, il vous est demandé soit de retirer. Cet amendement ou et à défaut un avis défavorable. La ministre mais ma vie. Je vais donc madame Ribet. je souris en écoutant votre argumentaire. Monsieur le rapporteur. Parce que vous voulez encourager les entreprises à embaucher des sapeurs-pompiers, mais en même temps moi je peux vous dire par expérience que cet été. Nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui travaillait dans un certain nombre d'entreprises n'ont pas pu être libéré parce que les entreprises n'ont pas voulu les libérer. Ils les ont libéré trois jours, quatre jours, 5 jours mais pas au-delà parce que c'était trop lourd et donc. Les sapeurs-pompiers. Ils ont pas d'autre solution que de prendre ça sur leurs congés personnels et au bout d'un moment ben ça commence à peser lourd. c'est un amendement essentiellement d'appel et je voudrais rappeler que dans la loi ma trace il y avait aussi un aspect pour favoriser. L'embauche de de sapeurs-pompiers et de dans dans les entreprises et on a rien vu venir. Donc l'objectif de cet amendement, c'était de mettre en alerte parce que vous pouvez bien avoir beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont employés dans le privé mais s'ils peuvent pas être libéré ben c'est c'est ça sert strictement à rien. Madame De Lattre. Oui merci madame la présidente. Je voudrais dire que je comprends complètement cet amendement d'appel parce que effectivement j'ai vécu les mêmes problématiques que que Laurence et nous avons eu beaucoup de témoignages en ce sens un amendement que nous aurions pu élargir chers collègues aux élus salariés puisque nous avons dû intervenir auprès. D'employeurs. Pour des maires qui était en train de de de d'évacuer leur population et devait être présent en tout cas il était fortement conseillé, qu'ils soient présents et heureusement qu'il était. Et nous avons eu des difficultés avec les employeurs donc. Il est normal que nous puissions relayé ici dans cet hémicycle. Ces dysfonctionnements et que nous essayons de trouver ensemble. Un moyen de de pouvoir avancer sur ces mobilisations. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. L'objectif de cet amendement consiste. En la mise en place d'un d'un plan transfrontalier de lutte opérationnel contre les incendies. De manière à coordonner la lutte contre les incendies entre les départements frontaliers et leurs homologues des pays voisins. En effet les pour aboutir à une une lutte efficace contre les incendies de forêt, il apparaît primordial de bâtir dans les territoires frontaliers des plans d'action opérationnelles permettant de s'entraider avec nos voisins pour aboutir à une lutte plus efficace. Face à un incendie majeur, le risque d'incendie ne connaît pas de frontières aussi cet amendement vise à inviter les collectivités mais vraiment à les inviter, je, j'insiste sur les termes et non pas les obliger. À mettre en place un plan et créer un dialogue opérationnel transfrontalier afin de mettre en place une synergie. Des organisations de défense contre l'incendie. Par là même un inventaire des moyens disponibles dans chaque département frontalier et leur équivalent dans le ou les pays voisins et de nature à cerner les éventuelles complémentarité matérielles et humaines et leurs limites dans la perspective d'un partenariat opérationnel ambitieux. J'étais je terminerai peut-être par un exemple extrêmement parlant, qui a eu lieu cet été pendant que nos. Véhicules d'incendie de secours étaient partis en renfort dans les Landes. Nous avons eu un incendie dans le dans la art et sans l'aide de nos amis suisses. C'est pas 10 hectares qui seraient partis en fumée, c'est 13.500. Voilà donc c'est c'est relativement parlant on a évité le pire je j'insiste par rapport à nos collègues rapporteurs on obligera, bien évidemment pas ni l'Allemagne ni la Suisse. Nous n'avons pas la compétence pour les obliger à faire quoi que ce soit simplement dans tout, dans toutes projet frontaliers ou transfrontaliers. Il faut qu'il ait un pays qui soit moteur et je vous invite simplement à mettre en commun les aventures qu'on aurait pu faire de part et d'autre, ça n'engage à rien de plus. Merci Oui, chers collègues. À la lire. D'une façon très précise l'objectif de votre amendement. Celui-ci est partagé sans aucun doute par tous les bancs de de l'hémicycle. Je ne peux cependant accordé un avis favorable à cet amendement qui imposerait la réalisation de ces plans transfrontières je cite aux autorités service compétents du ou des pays limitrophes. Puisque votre amendement soumet ses plans alors à. Et à leur coopération. Il est donc pas envisageable d'inscrire de tels plans dans le code forestier qui ne s'applique que sur notre territoire. Le territoire national français la bonne échelle serait soit une initiative spontanée. De la part des services concernés par des coopérations. Qui peuvent être tout à fait il. Il y a pensé on on a des coopérations entre SDIS. À l'intérieur de de même région dont pourrait tout à fait l'imaginer. Soit une initiative portée à l'échelle, bilatérale ou européenne en l'état, c'est un avis défavorable. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, en effet. De l'un des. Explications de vote de monsieur le rapporteur ou de, ou d'avis. Vous dire qu'en fait votre préoccupation. est déjà prise en compte dans le cas des dispositifs de gestion de crise existant. Il y a déjà de la contractualisation entre différents pays sur le sujet de la lutte contre les incendies. Donc la Commission européenne en collaboration avec les administrations nationales concernées a mis en oeuvre le système européen d'information sur les feux de forêt ce système accessible en ligne est un système d'information géographique qui fournit des informations en temps réel sur les feux de forêt et le régime en Europe. Ce dispositif a été créé afin de soutenir les services chargés de la protection des forêts contre les incendies dans l'UE et les pays voisins et puis de fournir aux services de la Commission européenne au Parlement européen des informations. Sur les feux de forêts en Europe donc pour les raisons invoquées. Nous vous demandons de bien vouloir le retirer. Sinon nous émettrons un avis défavorable mais je m'engage dans le cas du travail que je conduis pour la mission transfrontalière à voir où nous avons des accords et où nous n'en avons pas et travailler sur les lieux sur lesquels nous n'en avons pas merci. Oui le 114, consiste lui à deux a précisé a demandé au gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Qui permettrait de déterminer justement dans les zones frontalières, donc ça revient un petit peu à ce que disait madame la ministre, à l'instant. Dans les zones frontalières où est-ce qu'il existe un un risque transfrontalier d'incendie majeur et il permettrait également d'évaluer pour chaque territoire identifier le niveau de risque. L'évolution envisagée le dresser un bilan des moyens existants et encore une fois, de mettre en en moyen et de mettre en oeuvre. comment les mettre en oeuvre pardon pour faire face à ce risque, il permettrait également de répertorier les coopérations transfrontalières existantes et il permettrait je fais rapide il permettrait d'identifier le cas échéant les territoires qui sont soumis à ces risques d'incendie. Celui-ci j'aimerais le maintenir, parce qu'il avait un avis favorable sauf erreur mais je vous laisse souffert. Il y avait un avis, excusez-moi. Comme c'est un rapport je n'avais pas anticipé qu'il aura un avis favorable mais je vais donner la parole aux rapporteurs. Non non oui non vous allez pas le voir madame la présidente. Non, non. Demande de rapport. Avis défavorable, chers collègues. Je vais laisser le soin. Travail. Merci Merci madame la présidente, et merci monsieur le rapporteur. Alors effectivement on est très solidaire sur. Le fait de de. Exigeait trop de rapport mais il est important, comme vous le soulignez Monsieur le Sénateur, d'approfondir l'organisation de la lutte transfrontalière comme je voulais proposer juste avant qu'il y ait une de nos solutions pour faire face à des épisodes intenses d'incendie mais aussi qui est un vecteur de solidarité à l'échelle européenne dans laquelle la France s'inscrit. Bien évidemment. Alors nous ne sommes pas opposés à rédiger un rapport au Parlement permettant de dresser un bilan de l'organisation de la lutte transfrontalière contre les incendies de forêt. Le bilan que vous souhaitez, demander au gouvernement devra s'appuyer sur le travail que devra réaliser au préalable. L'Union européenne dans le cadre de l'analyse du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Voilà donc j'émets. Un avis favorable à votre amendement. Monsieur le sénateur. Bien nous avons donc un amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour.

Madame la présidente. Merci. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Donc l'objet de cet amendement et la reconnaissance de la dangerosité du métier des personnels navigants de la sécurité civile le présent amendement tend à reconnaître l'Exposition danger des personnels navigants de la sécurité civile pilote, copilote mécanicien. Opérateur de bord et personnel navigant cabine durant l'exercice de leur métier, la nation a reconnu le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers professionnels depuis 2004 dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile. Le gouvernement propose aujourd'hui d'étendre cette reconnaissance au personnel navigant qui risquent leur vie à chaque vol pour sauver celle de nos concitoyens ou protéger nos espaces naturels. Cette reconnaissance symbolique s'inscrit dans une volonté d'amélioration du statut des personnels navigants de la sécurité civile alors même qu'ils sont confrontés à des phénomènes d'ampleur durant les saisons de feux de forêt que le territoire national connaît désormais chaque année et que les interventions de secours à personnes se multiplient sur tout le territoire national. Je vous remercie. Ce sera un avis favorable. La reconnaissance par la loi de la dangerosité des fonctions de de des métiers que Madame la Ministre vient d'évoquer une façon de rendre hommage à ces personnels alors que les accidents mortels ne sont malheureusement pas rares. Le dernier remonte à l'été 2019. Nous ne pouvons donc donné un avis favorable à cet amendement qui je l'espère fera consensus parmi parmi nos bancs. Eh bien je vais mettre voix cet amendement sans humide qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour.

Merci madame la présidente. Le 11 octobre dernier lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. S'était alors engagée à étudier l'opportunité de la création d'une seconde base pour les canadairs et autres et honnête de la sécurité civile. En plus de celle de Nîmes afin de concrétiser les engagements du gouvernement cet amendement vise à réaliser une étude de faisabilité pour l'installation de cette seconde de base. Tous les acteurs sont unanimes, plus le feu et repérer et traiter rapidement, plus les chances l'essence de l'éteindre sont renforcés. On de l'Exposition colossal de nos forêts de l'ouest de la France au risque incendie. Cette base est essentiel R permettra à la sécurité civile n'intervenir au plus vite et au plus près des, des, pas de feu. merci madame la présidente. Les feux qui ont frappé la Gironde cet été ont en effet mis en évidence la nécessité d'une meilleure couverture du territoire. Par les moyens aériens de lutte anti-incendie qui relèvent de l'État puisque les moyens aériens sont de la compétence de l'État. Toutefois l'opportunité d'ouvrir cette nouvelle base une nouvelle base. Au-delà de celles qui existent aujourd'hui à Nîmes, ne constitue pas une évidence plusieurs acteurs de la lutte contre les estime que l'ouverture d'une 2ème base. Impliquerait une dispersion des moyens aériens, rendant de fait plus délicat, leur capacité de projection et leur coordination ainsi qu'une multiplication des coûts de maintenance des appareils. Je souhaiterais donc entendre l'avis du gouvernement sur cet amendement et sur les pistes qu'il a identifié pour améliorer la couverture du territoire par nos moyens aériens de lutte contre les feux de forêt. Merci madame la présidente. Et. Madame la sénatrice de Paris. On joue c'est très engagé sur ce sujet. De la lutte contre les feux de forêt votre amendement nous donne l'opportunité de vous redire l'engagement du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a mené une étude pour la création d'une seconde base de sécurité civile. Les services sont mobilisés dans ce sens il travaille activement à ce sujet pour faire émerger des pays viable en réponse à ce chantier d'ampleur. Vous serez donc tenu informé des évolutions et de l'avancement de ces travaux, la création d'une seconde base de sécurité civile nécessite des moyens et des infrastructures conséquente. Pour exemple la base de sécurité civile. Nîmes a été créé en 2017 avec un investissement majeur de près de 17 millions d'euros en complément d'installations aéronautiques déjà existantes. Elle exige également un travail avec nos partenaires industriels qui réalise la maintenance de nos aéronefs dans l'attente de la réalisation de cette étude pour la création d'une seconde base les implantations de détachements temporaires opérationnel d'aéronefs de la sécurité civile sur le territoire national sont déjà une réalité aujourd'hui le ministère de l'intérieur des Outre-mer, être en capacité d'armer des détachements sur tout le territoire en tant que de besoin, comme ce fut le cas à Bordeaux durant l'été grâce à son réseau de 22. Drôme. La souplesse de l'organisation opérationnelle actuel permet de faire face aux enjeux et de projeter des détachements en fonction de l'analyse des risques et des besoins. Nous tenons à préciser que le renouvellement de la flotte actuelle des hélicoptères de la sécurité civile et son accroissement à 40 appareils. Mesure portées dans le cas de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur vont permettre à la sécurité civile de réinvestir le Champ d'émission de bombardiers d'eau avec des appareils plus puissants et mieux équipés que ceux actuellement détenus avec la location d'hélicoptères bombardiers d'eau lourds. Cette mesure aura pour conséquence de disposer d'une capacité bombardiers d'eau sur de multiples bases réparties sur tout le territoire et en particulier dans le Sud-Ouest. Donc votre amendement est tout à fait. Madame la sénatrice. En conséquence de quoi, comme monsieur le rapporteur. Je vous demande de bien vouloir le retirer. Alors monsieur le rapporteur. Maintenant que vous avez entendu la ministre. Quel est votre avis.

Cette éventualité d'une création d'une nouvelle base parce que d'autres territoires. Ont également fait des propositions, je ne suis pas le porte-, parole de de territoires alors pas la Normandie hein je vous rassure, on est on n'est Demande d'une étude de faisabilité pour la création d'une nouvelle base aérienne de la sécurité civile. Est-ce que Madame de Marco. Dans votre. Comment dire amendement. Vous parlez bien du Sud-Ouest de la France.

Pour la création d'une nouvelle base aérienne sans donner un territoire. Préalablement arrêtée là, vous demandez une étude de faisabilité pour la création d'une base aérienne dans le Sud-Ouest de la France, c'est quand même pas la même chose. Donc j'aurais tendance à rejoindre. L'avis du gouvernement. Et d'émettre un avis défavorable sur la demande que vous faites encore une fois je la reformule j'ai sous les yeux le, le, le projet d'amendement étude de faisabilité pour la création d'une base aérienne de la sécurité civile, dans le Sud-Ouest de la France. Il aurait été tout autrement. Et la position. De de la commission aurait été tout autre. Il s'il avait s'agit d'une demande d'une étude d'opportunité pour la création d'une nouvelle base aérienne de sécurité civile, sans préciser le territoire.

Nîmes devenait une base européenne, sécurité des civils et monsieur le ministre a dit que il était possible d'envisager une seconde de base mais ici-même et je pense que le. le rapport fait froid que il a dit qu'elle serait plutôt au nord de la Loire qu'au sud de la Loire a priori son avis qui donnait et que donc c'est vrai que je reconnais et je rejoins. L'honorable rapporteur de maîtres que dans votre amendement dans le Sud-Ouest. Je pense que déjà ça limite trop vous auriez mis. Une seconde base ça aurait été peut-être plus acceptable pour pour tout le monde et puis ma chère collègue peut être ce soir, on a beaucoup de sagesse dans cet hémicycle. Je crois qu'il serait intéressant. Pour vous de Marco comme d'autres de venir visiter la base écrire des civils et de Nîmes. a rencontré le personnel et vous verrez que. Le personnel moi je les ai rencontrés pendant 3h. D'abord ce sont des gens. Charmants très professionnel et qui vous expliquent que ce que l'on peut comprendre lorsqu'on n'a pas cette information. Un Canadair. Rwanda, ça ne se met pas comme cela. Un Canadair. Il faut qu'il y ait des Ethan ou de la mère qui puissent pouvoir piocher eau d'Dash, il faut un aéroport avec certaines conditions et donc vous avez une cartographie à la base à scruter qui montre là où le Canadair Dash je pourrais aller et je pense qu'avant de déposer type d'amendements.

Oui merci madame président moins un ministre monsieur le rapporteur, chers collègues. Effectivement nous avons eu ce débat sur le texte de la loi Lopmi. J'avais d'ailleurs déposé un amendement que j'ai retiré. Suite à l'explication et l'engagement du ministre de l'Intérieur Darmanin. Qui et je rejoins complètement notre rapporteur on n'était pas sur une autre base. On était sur une architecture. De la base de Nîmes. Qui était le coeur central pour notre pays. Et d'avoir répartis sur le territoire pour traiter à la fois le Sud-Ouest. L'Ouest et l'Est de la France et je rejoins le débat qu'on avait sur transfrontalier parce qu'effectivement on a une zone. Et notamment on avait la base de de Mirecourt qui est équipé qui il y a eu des tests d'ailleurs qui est équipé pour le. Les recevoir dépendant de Nîmes, il n'était pas question de refaire et et moi ça me pose problème de limiter à une. C'est pas possible parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le risque forestier. Et l'ampleur l'intervention la plus rapide est nécessaire elle nécessaire à la fois pour le Sud-Ouest est nécessaire aussi, on l'a vu dans, dans l'ouest de la France et est nécessaire aussi, dans l'est de la France donc. Je rejoins notre rapporteur. Pour cette raison, moi je ne veux pas voter cet amendement là c'est il est trop restrictif et il est. Restrictif surtout par rapport aux engagements du ministre de l'Intérieur qui avait été pris dans le débat et c'est comme cela d'ailleurs que je vais retirer mon amendement compte tenu qu'. Il y avait un engagement très clair du ministre sur cet aspect des choses. Oui merci madame la présidente, mes chers collègues, effectivement. Je dirais, dans le sens du du rapporteur, et pourtant je suis girondine. Mais je pense qu'il est malheureux effectivement que nous ayons que vous ayez rajouter chers collègues le Sud-Ouest même si je peux le comprendre. Mais effectivement, nous avons un réchauffement climatique. Nous avons déjà une base dans le sud. Et si nous en obtenant une de plus dans, dans le Sud-Ouest, nécessairement, il en faudra une 3ème voire une 4ème. Selon les les cadrans dans en France entière, on l'a dit, c'est quand même un coût conséquent moi je me suis battu pour le prépositionnement. Le ministre a donné plutôt un avis positif sur ce prépositionnement c'est ce qu'il devait confirmer en annonce lors de son déplacement qu'il a dû annuler. Il y a quelques jours. Moi voilà je je pense que un prépositionnement. Avec la base de Nîmes. Et aujourd'hui, plus réaliste, plus pragmatique et s'il devait y avoir effectivement 3ème 4ème base. Ce sont des fonds que l'on ne mettrait pas sur du matériel qui qui nous est indispensable d'avoir des avions supplémentaires

en tout cas sur le le scrutin public. Je ne peux pas. Vous l'avez compris, voter pour. Compte tenu de, de la rédaction que vous proposez. Merci. Oui, je vous remercie donc pour ma part je ne suis pas dans les confidences, je ne sais pas ce que les 3 ministres qu'il se il se déplacer dernièrement en Gironde. Devait annoncer. Toujours est-il que je rappelle donc. Ce n'est pour l'instant qu'une étude de préfiguration mais je vous ai pas dit qu'on allait implanter dans le Sud-Ouest, une base. Non non non alors je veux bien retirer. Dans l'amendement le terme de Sud-Ouest. Mais vous vous emballez beaucoup. Je demande simplement qu'il y ait une une étude d'opportune et de la crise pour la création d'une base aérienne de la sécurité civile. En France, alors dans ces conditions. Peut-être que vous pourriez voter cet amendement. Madame. Harribey. OK. Monsieur gay. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Moi je n'ai aucun intérêt en Gironde, même si c'est un très beau département. Que je connais bien. peu importe, moi je pense que c'est mieux. La rédaction sur l'opportunité mais la question fondamentale c'est qu'aujourd'hui on a 21 avions de 35 hélicoptères. On nous a dit. Après la sécheresse et les gros incendie on va investir. Bien sûr, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais. Quelle est la direction vers laquelle on va et à quelle échéance. Quand on sait qu'on va avoir des nouveaux bombardiers quand c'est que nous aurons des nouveaux le code terre. Est-ce que par exemple depuis les incendies que nous avons connu, il faudra du personnel aussi former. Et ça se trouve pas là aussi en quelques semaines. Parce que vous pouvez avoir après avoir le bombardier le Canadair, l'hélicoptère mais après il faut pouvoir évidemment le. Le manoeuvrer et donc ça pour l'instant on a du mal à voir les investissements qui sont mis. Et malheureusement la sécheresse que nous connaissons en plein coeur de l'hiver nous font craindre et personne. Ici ne le souhaite mais encore un été extrêmement jour et potentiellement avec des méga feu et malheureusement vu le dérèglement climatique. C'est une question qui va se poser. Aujourd'hui, dans le Sud-Ouest, mais un peu partout, j'ai envie de dire, en France, donc y compris il faudra regarder comment on prédisposent l'ensemble du dispositif sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ça les questions qui à un moment donné qu'il va donc falloir vous poser et apporter des réponses. Ce que nous pensons que ça se réglera pas en quelques semaines. Mais par contre il ne faut pas que l'été prochain on nous dise ah comme ça, on n'avait pas le matériel mais vous inquiétez pas, ça va arriver, puis 2024 puis 2025 plus 2026. Il faut nous dire dès maintenant, on veut auprès recruter et on veut former et voilà vers là où on va mettre l'argent pour recruter et former et avoir du matériel, je vous remercie madame la présidente. Monsieur Bourgi. Voilà la présidente Madame la Ministre je voudrais prolonger le propos de notre collègue. Gay pour dire qu'effectivement le débat que nous avons ce soir me rappelle furieusement les débats que nous avons eu il y a quelques mois et à plusieurs occasions avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pendant très longtemps la doctrine de la France en matière de lutte contre les feux de forêt reposé sur la coopération européenne à la solidarité européenne malheureusement avec le changement climatique. La France comme les pays voisins du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la Grèce parfois peuvent connaître des épisodes particulièrement violent de manière concomitante, donc cette solidarité qui s'exprimait par le passé s'exprime beaucoup moins de manière efficiente. Donc il faut demander la solidarité de pays européens qui sont beaucoup plus éloignés de notre pays. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur avait évoqué plusieurs pistes, à savoir une coopération, une coordination européenne pour commander faire une commande groupée de Canadair par exemple aujourd'hui nous n'avons pas le début des éléments de réponse que nous attendons de sa part avait été évoqué la possibilité de faire de Nîmes. Le lieu central pour le reconditionnement la révision la réparation. des Canadair et les Dash et peut être imaginé qu'il puisse y avoir des prêts prise seulement ailleurs dans la dans notre pays là aussi une étude prospective devait avoir lieu pour voir ce qu'il était utile de faire parce que le ministre il n'avait pas les réponses à l'époque et je le conçois parfaitement aujourd'hui j'ai le sentiment que nous entamons bientôt la 2ème campagne de feux de forêt après celle de l'été dernier et des éléments de réponse que nous attendions depuis plusieurs mois ne sont toujours pas arrivés. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait peut-être bon qu'on se hâte pour répondre à ces questions qui restent prégnante dans nos territoires et auprès de la population et auprès des forces de sécurité civile, il nous faut vraiment apporter ces réponses. Ne pas donner le sentiment que nous procrastination. Merci, madame la Ministre. Non pour conforter Merci madame la présidente, avait proposé à l'unanimité des de commission de l'aménagement du territoire et des affaires économiques 70 recommandations dont celle qui porte le chiffre 60 je je vous je vous la lis étudier l'opportunité. De créer une 2ème base aérienne de la sécurité civile pour plus de rapidité dans la mobilisation des moyens de lutte. Donc on parlait d'opportunité et on ne parlez surtout pas de signe particulier sur sur le territoire national recommandations 60. Madame la Ministre. Merci. Madame la présidente. Je voudrais juste. M'adresser à Madame la sénatrice de. vous je conclus en vous disant que votre amendement est satisfait, je les, je vous voyez. Peut être ne ne ne pas être en adhésion avec mes propos. Mais votre objet c'est une étude de faisabilité pour la création d'une 2ème base de sécurité civile, dans le Sud-Ouest. Moi je vous ai confirmé. L'engagement du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a mené une étude pour la création d'une seconde base de sécurité civile évidemment pas dans le Sud-Ouest et ça a été rappelé par le sénateur quoi que je remercie. Cet engagement à conduire une étude elle est totale. Donc quand je vous dis simplement, elle n'est pas encore fait par contre un certain nombre d'éléments que j'ai développé, que je ne vais pas vous relire monde que certains nombres d'actions et d'ailleurs la sénatrice Delattre a indiqué. Sauf dans le Sud-Ouest, dans mon texte. Moi j'ai pas la dimension Sud-Ouest dans mon texte et donc je disais que la sénatrice Lattre a indiqué que. Il y avait une réflexion autour d'un prépositionnement. D'avions, d'hélicoptères. Et ça fait partie de tout l'arsenal sur lequel le ministre de l'Intérieur est en train de travailler. Je vous ai indiqué. L'augmentation de la flotte je vous ai parlé de location d'hélicoptères de renouvellement d'hélicoptères. en fait le ministre de l'Intérieur, il est dans la continuité de ce qu'il vous a dit, le travail sur le fait que la base de Nîmes devienne une base européenne cela avance bien, il m'a demandé de le représenter dans une rencontre avec le ministre grec. De la gestion de crise et que j'ai reçu en son nom et avec lequel nous allons porter le développement de cette base de Nîmes comme étant une base européenne. Donc oui aujourd'hui on n'est pas en mesure. De vous faire partager les conclusions d'un rapport mais par contre le fait que l'étude hé bien le ministre de l'Intérieur, soit engager et il travaille. C'est une réalité, l'engagement que j'ai pris aujourd'hui de vous faire partager les avancements de cette étude aussi et la création de cette seconde base de sécurité. Je vous ai simplement donner des montants comme 17 millions puis je salue les propos de monsieur qui indique à quel point. Les enjeux sont importants en termes de formation, donc tout ça pour dire que ça n'est pas quelque chose de simple, mais que je pense que ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une étude de faisabilité, hé bien elle est tout à fait satisfaite. Voilà donc c'est pour cela que je vous appelle à bien vouloir retirer aujourd'hui. Aujourd'hui dans le cadre de la réflexion que nous conduisons aujourd'hui. Votre proposition est votre amendement. Merci merci madame la présidente dans c'était juste et ce que ma, ma collègue. Monique de Marco là la expédie tout à l'heure, c'est qu'on on a on a entendu les différentes remarques qui ont été faites et donc on propose de réécrire l'amendement et de juste supprimer la localisation. Et donc d'avoir le gouvernement réalise une étude de faisabilité pour la création d'une base aérienne. De la sécurité civile. Il me semble que c'est important que cet amendement puisse être voté dans ces termes là sans localisation et notamment moi j'entends ce que ce que dit ce que, ce qu'a expliqué Madame Madame la Ministre mais c'est vrai que si s'est engagé peut-être je sais pas mais en tout cas ça me ça permet que ça soit. Dans la loi et qu'on ait cette réflexion sur l'opportunité d'une nouvelle d'une nouvelle base aérienne effectivement quelle que soit la localisation. Je pense que, a priori c'est ce qui était partagée par tout le monde et donc ça me paraît important qu'on puisse. Réécrire ce cet amendement et du coup de le voter. Merci. Monsieur le président Gontard. Madame de Marco. Si vous m'autorisez, je vous propose la rédaction suivante le gouvernement réalise une étude de faisabilité pour la création d'une nouvelle.

de avis j'essaie de trouver une rédaction qui soit à peu près cohérente par rapport à la discussion qui a été conduite. Il faut bien dire qu'elle est nouvelle et l'étude et ce n'est qu'une étude de faisabilité. Voilà. Bon si Madame de Marco qui d'autres. L'autrice de l'amendement. Accepte cette rédaction. Je vous propose de la retenir, merci et donc. Je rappelle pour autant que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement est défavorable et le scrutin. Cela. Alors est-ce que la commission change d'avis avec la nouvelle rédaction. Enfin du moins ce que le rapporteur change d'avis. Alors. Nous, nous avons parlé d'une étude non pas de faisabilité mais d'opportunité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc la la la la recommandation 60 parler d'une étude d'opportunité pour la création d'une éventuelle 2ème base aérienne. Bien donc l'avis de la commission reste défavorable amendement reste tels que Madame de. En mettant opportunité ça serait possible que nous revoyons donc la rédaction.

C'est pas une opportunité à, à l'heure qu'il est effectivement il y a eu des explications du rapporteur il y a eu des explications de Madame la ministre il y a eu des engagements du ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on ne va pas refaire l'amendement complètement ce soir. Ça me paraît pas tout à fait opportun. Donc. On maintient étude de faisabilité. Si je comprends bien. Et on enlève Sud-Ouest. Vous êtes d'accord monsieur le président. Voilà on enlève Sud-Ouest le gouvernement réalise une étude de faisabilité pour la création d'une nouvelle base aérienne de la sécurité civile. Voilà l'amendement telle qui sort des discussions et donc le scrutin. Donc, les avis sont défavorables de la commission du gouvernement et le scrutin est ouvert.

ouvert. Ça ne demande à voter. Le scrutin est clos. 343, 329 pour 90 contre 239, le Sénat n'a pas adopté bien il nous reste. Je crois cinq amendements. À examiner. Est ce qu'on pourrait être d'accord pour. Le faire à un rythme un peu soutenu. Merci. Donc. L'amendement 111. Monsieur bus. Voilà. Oui merci madame la présidente à l'article 34 10 propose de sécuriser juridiquement l'emploi des coupes tactique lors des opérations de lutte comme cela a été le cas au cours de l'été 2022 dans les Landes et en Gironde. L'heure est texte fait après ces incendies a montré tout l'intérêt de ce dispositif de création de lignes d'appui à la lutte pendant le sinistre mais aussi des problèmes générés par celui-ci. L'amendement proposé vise donc à compléter l'article 34 bis hein, sécurisant juridiquement la prise de décision et en assurant grâce à la réquisition un juste dédommagement des entreprises qui réaliseront les travaux et des propriétaires de terrains qui verront leur leur. Transformées en ligne d'appui à la lutte. Qui est contre qui s'abstient est adopté l'article 34 bis inquiet pour qui est contre qui s'abstient il est adopté. L'amendement 103 Madame la Ministre. Merci madame la présidente article. 35, amendement 103, nous proposons la suppression des conditions énoncées dans l'article 35 concernant l'attribution des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois. Ces précisions ne sont en effet pas permis. Sinon, dans la mesure où le code forestier énonce déjà clairement elle 121 tirer hein et de manière plus complète au regard de la multi-fonctionnalité des forêts et les différents enjeux les objectifs poursuivis en matière de politique forestière qui s'applique par construction aux aide au reboisement. Par ailleurs, le code forestier prévoit déjà Howell 121 tirer six que le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts subordonnée à l'existence d'un document de gestion durable qui est agrée par l'État sur la base de documents d'orientation sylvicoles justement. En cours de révision et prenant pleinement en compte les enjeux de résilience et l'adaptation des forêts au changement climatique. Néanmoins il est clair qu'il convient de compléter cet article L. 121 tirer hein. En ce qui concerne la politique de lutte contre les incendies. Sur ce dernier point, je vous propose d'ailleurs dans un nouvel article d'intégrer cette mention spécifique. Je vous remercie.

Pardon, juste pour dire quand même que cet amendement que je vous propose adopté vise à préciser renforcer la proposition concernant de la vice-. Diversification des essences. OK il y en a que deux. Alors, allons-y maintenant madame la rapporteure. La présidente. Alors les amendements, 97 et 127 nous semble aller un peu trop loin en détaillant précisément dans la loi, les conditions concrètes de diversification pouvant donner accès aux aides publiques en dessous et au-dessus de certains somme il nous semble important de poser le principe de la diversification dans la loi, c'est ce que nous faisons, mais nous sommes tout aussi important de préserver les marges de manoeuvre des propriétaires et des gestionnaires forestiers dans la déclinaison de ce principe sur l'ensemble des territoires. En outre, et compte tenu des réserves exprimées par le le gouvernement. Il nous sommes mes chers collègues, ce serait délicat d'aller encore plus loin pour la suite de la navette et pour pour l'avenir de la PPL, s'agissant de l'amendement du gouvernement qui renvoie donc aux objectifs très généraux de la politique forestière définie à l'article 121 Ces dispositions Madame la Ministre toute force juridique et toute portée concrète au dispositif que nous avons mis en oeuvre dans cette PPL et qui vise à ajuster notre action à l'intensité. Des feux extrêmes auxquelles nous sommes confrontés dans une urgence. à quelques mois de la saison des incendies alors qu'on voit déjà des incendies naître. Sur tout le territoire. Donc l'enjeu, la prévention et la lutte contre les incendies de forêt ne peut s'accommoder Miss ils vont pas si l'expression d'un droit mou. Nous partageons bien sûr vous l'avez dit, l'objectif de ne pas imposer des pratiques sylvicoles qui serait descendante et qui serait excessive. C'est pour savoir que nous renvoyons au règlement de la définition concrète de ces principes, donc je vous proposerai. Face à ces trois amendements qui sont aux antipodes. Hé bien d'adopter la proposition de sagesse de la commission. madame la Ministre, quel est votre avis sur les deux amendements identiques, 97 et 127. Même avis que la commission sur. L'amendement 97 et 127. Je vais donc commencer par mettre aux voix l'amendement 103 amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui contre qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement. Les 2 amendements identiques double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés article 35 et pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 128 Madame de Marco. Très rapidement cet amendement propose reconnaître le rôle des associations syndicales de défense des pour et contre un incendie dans la promotion de l'assurance des parcelles face aux risques d'incendie et de tempête.

cela passe par la loi qui elle compte qui s'abstient il est adopté. Article 37 même vote même votre article 38 nous avons une demande de parole de madame la présidente Delattre. Oui merci madame la présidente. J'ai trouvé cet endroit pour poser cette question à madame la ministre. Madame la ministre, vous veniez début août. À Kenzo et je vous avez fait part de la demande des, des communes. De pouvoir utiliser la DETR la le le Fonds Vert. Pour prendre en charge. Les dégâts des incendies. Sur des bâtiments communaux sur les voiries communales. Vous m'aviez indiqué que vous alliez regarder et avec les ministres concernés. Je vous ai posé cette question en discussion PLF pareil vous m'avez dit que vous alliez regarder. Je n'ai pas vu. Dans. Le règlement DETR et décide de la Gironde l'opportunité. Ouverte par le préfet de prendre en charge. Ces surcoûts liés à ces incendies par les collectivités donc sur DETR décide il me reste un espoir, c'est sur le fond Vert. Puisque nous n'avons pas encore eu l'arbitrage du du préfet. Et d'indications en la matière. Donc voilà je voulais vous poser cette question ce soir parce que beaucoup de communes sinistrées sont en attente de cette possibilité. Merci. Merci madame la ministre. 152. C'est la levée du gage Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Et. Mesdames, et messieurs les sénateurs, donc par cet amendement de suppression. Le gouvernement souhaitait tout simplement levez le gage madame la sénatrice de être. En fait, y a aucun rapport entre. Est ce que vous vouliez répondre à Madame De Lattre. Oui. Merci. Merci madame la présidente. C'est c'est effectivement un amendement de suppression de l'article 38 qui gager la PPL alors cet amendement étant arrivé de façon plutôt tardive. Je je m'exprimer. Oui je l'ai là. Je m'explique, je la commission n'a pas pu se réunir pour se prononcer cet amendement donc je m'exprimerai. À titre personnel et je donnerai un avis à titre personnel. Mais je tiens à préciser que je vois dans cet amendement, un signe de soutien du gouvernement. Sur cette PPL qui augure d'une suite très prochaine de la navette. Et donc personnellement j'émettrai un avis favorable sur cet amendement, merci. Je vois plus. Bien alors je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable et personnel du rapporteur. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Et donc l'article est supprimé. Voilà et je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des explications de vote. Non c'est très raisonnable. Voilà Voilà donc. Qui est pour la proposition loi. Qui est contre. Je n'en vois pas qui s'abstient. Il n'en a pas non plus la proposition note pas adopté à l'unanimité. Mes chers collègues. La prochaine séance aura lieu ce mercredi 5 avril à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement et la séance est levée.